mes chers collègues, à vous assurer que vous disposez bien de votre carte de vote et à vérifier que celle-ci fonctionne correctement

Or le rapport de la Cour des comptes montre que non seulement il n'y a pas d'économies, mais qu'en fait les grandes régions coûtent cher ! Bien sûr ! C'est une véritable aberration ! Je prendrai l'exemple du Grand Est,

Étant élue régionale du trop grand Grand Est et habitant dans la Marne, pour aller au chef-lieu, à Strasbourg, c'est 332 kilomètres,

Ainsi, nous aurons à débattre très prochainement du projet de loi de finances, qui, force est de le constater, ne répondra pas aux besoins de financement des collectivités territoriales.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, qu'il est difficile, en France, d'échapper à la tentation de concentrer, de centraliser et d'uniformiser tout ce qui relève du politique et de l'administration Cette obsession, qui remonte au moins à Philippe le Bel, a été partagée par tous ses successeurs et, contrairement à ce que l'on croit parfois, elle s'est encore renforcée sous la Révolution, comme l'a magistralement démontré Tocqueville. En 1800, Chaptal expliquait à l'Assemblée nationale : « Le préfet transmet les ordres au sous-préfet, celui-ci aux maires des villes, bourgs et villages, de manière que la chaîne d'exécution descend sans interruption du ministre à l'administré, et transmet la loi et les ordres du Gouvernement jusqu'aux dernières ramifications de l'ordre social avec la rapidité du fluide électrique. Cette description nous fait sourire aujourd'hui, quarante ans après les premières lois de décentralisation. Mais, si l'on remplace dans ce texte le politique par l'administratif, et les ministres, préfets et sous-préfets par les experts, technocrates et bureaucrates, sommes-nous encore certains que les choses ont autant changé que cela ? C'est bien l'un des sujets qui nous réunit aujourd'hui et cette loi NOTRe et sa rigidité éloignée des spécificités locales, véritable lit de Procuste dont nous cherchons à scier les barreaux, Un de nos collègues me disait que ce projet de loi était celui des frustrés de la loi NOTRe. Vous nous dites, monsieur le ministre, qu'il vise à gommer les irritants de cette loi, que l'on pourrait résumer d'une formule : « Chérie, j'ai rétréci les maires ! Nous ne pouvons qu'être d'accord avec votre intention. répond selon moi à un deuxième objectif, mais je ne suis pas certain que vous l'admettriez publiquement. Il s'agit d'obtenir que les maires vous pardonnent.

bien ! ... mais à tous les gouvernements et à toutes les assemblées responsables des multiples lois de décentralisation et de déconcentration mises en oeuvre depuis des années, qui n'ont souvent apporté que des réponses cosmétiques aux besoins des collectivités, quand elles n'ont pas elles-mêmes aggravé les problèmes. est résulté des territoires en grande difficulté, auxquels on demande pourtant de réduire leurs budgets, des élus qui ne savent plus quoi faire pour ne pas laisser dépérir leurs villages, des communes rurales sans moyens humains et financiers pour soutenir le lien social et économique. La liste des difficultés est impressionnante : classes fermées, centres-bourgs qui perdent leurs commerces, services publics menacés, finances locales asphyxiées, déserts médicaux, fracture numérique ... Chacun d'entre nous sait cela. Comme dans les romans ou les films qui se terminent bien, vous vous présentez devant nous, monsieur le ministre, dans le rôle du rédempteur. Je ne sais si cette rédemption mènera au salut, mais, comme vous l'avez constaté tout au long de ces débats, le Sénat non seulement ne s'y est pas opposé, mais a souhaité y participer activement. Je voudrais, à cet instant, féliciter nos deux rapporteurs, Françoise Gatel et Mathieu Darnaud, ainsi que le président Philippe Bas, qui n'ont pas ménagé leur peine. Vous souhaitez tout d'abord renforcer le rôle des maires au sein des intercommunalités. Le Sénat a voulu consolider la place des communes et des maires dans le fonctionnement des EPCI, assouplir la répartition des compétences entre les échelons territoriaux et faciliter le fonctionnement des conseils municipaux dans les petites communes. Vous souhaitez renforcer les pouvoirs de police du maire. Le Sénat y a ajouté les mesures de nature législative de son plan d'action pour la sécurité des maires. Vous souhaitez simplifier l'exercice quotidien des compétences de la commune par les maires. Le Sénat a voulu étendre leurs pouvoirs et leur information. Enfin, vous souhaitez renforcer les droits des élus locaux. Le Sénat vous accompagne, en insistant plus particulièrement sur les possibilités de formation et les conditions d'exercice de leur mandat. Cette loi constituera-t-elle une révolution ? Non, et d'ailleurs personne ne le demandait. Car si les maires sont très critiques des lois qui régissent aujourd'hui leurs compétences et leur statut, il y a une chose qu'ils craignent plus que tout-ils ne cessent de nous le dire -, c'est un énième bouleversement qui ajouterait à ces défauts celui de l'instabilité législative, véritable plaie de notre pays. Ce projet de loi constitue une étape. Le Gouvernement nous annonce qu'il sera suivi l'an prochain d'un texte portant sur la décentralisation, la déconcentration et la différenciation. Le Sénat, chambre des territoires, l'examinera et l'enrichira avec la même rigueur et le même sérieux que pour le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie Le travail sera-t-il alors abouti ? Pas tout à fait, car il restera un immense chantier qu'aucun gouvernement n'a osé pour l'heure mener à bien, ce qui est pourtant l'une des conditions pour une bonne administration des collectivités : je veux parler de la réforme courageuse de la fonction publique et la définition d'un vrai statut de l'élu. Il nous reste donc beaucoup de chemin à parcourir ; nous n'en sommes qu'au début, mais Aristote disait que « le commencement est la moitié du tout ». Soyons optimistes, et considérons donc que nous avons ensemble fait un pas en avant significatif. Notre groupe votera ce projet de loi tel qu'amendé par nos travaux. La parole est

ce projet de loi, dont nous venons de terminer l'examen après quarante-cinq heures de séance publique, porte l'ambition de favoriser l'engagement dans la vie locale et la proximité dans l'action publique : tout un programme !

Quand les uns sont les sentinelles de la démocratie, les autres sont les citadelles de la République, et, dans un pays où les corps intermédiaires sont affaiblis, le pouvoir exécutif s'est naturellement tourné vers les représentants les plus proches du terrain pour recoudre le tissu social.

grande », une petite République au service, voire au secours, de la grande. C'est pour cela, mes chers collègues, que, dans cette situation, le Sénat n'a pas voulu, ne veut pas d'un rendez-vous manqué- d'un nouveau rendez-vous manqué, Avec la méthode et la constance qu'on lui connaît, la Haute Assemblée a donc voulu enrichir le texte en se fondant sur les travaux menés ces derniers mois notamment par la commission des lois et la délégation aux collectivités territoriales, qui ont été souvent soumis au vote du Sénat et si peu souvent repris à l'Assemblée nationale ... Je veux à cet instant féliciter nos rapporteurs, Françoise Gatel et Mathieu Darnaud, qui se sont imprégnés du texte du Gouvernement, en ont partagé les finalités et ont su nous en proposer une mouture fiable et enrichie. Ils l'ont fait en tentant d'éviter trois écueils la proximité des élections municipales, qui auront lieu dans cinq mois ; la diversité des sujets abordés, tant il est nécessaire, pour le législateur, d'intervenir en urgence dans des domaines où les collectivités sont en souffrance l'articulation avec un texte futur dont les contours restent incertains et dont on attend un nouveau souffle pour la décentralisation, une décentralisation de « nouvelle génération Notre groupe, fidèle à ce qu'il est, décentralisateur et girondin, a pris toute sa part à ce travail. À de nombreuses reprises, nous avons été suivis par des collègues siégeant qu'il s'agisse de mesures techniques de bon sens ou attendues, ou encore de vrais progrès pour nos communes et nos intercommunalités. J'en rends grâce aux nombreux collègues du groupe présents tout au long de l'examen du projet de loi, et en particulier à mes collègues désignés chefs de file avec moi sur ce texte, Laurent Lafon et Jean-Marie Mizzon.

relayés en séance par le président Philippe Bas alors que leurs amendements n'avaient pas passé les fourches caudines de l'article 40. Je ne peux pas ne pas relayer auprès de vous, monsieur le ministre, les inquiétudes de nos collègues polynésiens, très attachés au principe d'égalité, sur l'applicabilité du titre IV à la Polynésie française. D'autres sujets brûlants mériteront d'être retravaillés : je pense notamment à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans les fonctions électives exécutives.

car c'est un sujet sur lequel les élus locaux nous interpellent constamment, surtout lorsqu'ils découvrent que l'intercommunalité pourra rendre des compétences à ses communes membres et que les conséquences en seront financièrement non négligeables si l'on ne corrige pas le mécanisme de l'intégration fiscale.

là deux exemples, très différents, qui démontrent, s'il le fallait, que l'accompagnement financier de l'État est le corolaire indispensable de nombreuses mesures figurant dans ce texte et qui risquent, sans cet accompagnement, de n'être que des annonces.

rien ne changera vraiment si la relation de l'État avec les collectivités locales n'est pas repensée fondamentalement et si les services de l'État dans les territoires ne font pas, eux aussi, leur. Hier encore,

patrie du quotidien de nos concitoyens, lesquels ont plus que jamais envie de retrouver le lien de proximité qui les unit

la start-up nation a découvert le principe de réalité, la démocratie locale et l'importance des maires, des conseillers municipaux, communautaires, départementaux ou régionaux : à la bonne heure ! Enfin ! Votre texte, monsieur Lecornu, était très ambitieux à en croire les déclarations d'intention. je remercie nos rapporteurs du travail qu'ils ont effectué. Oui, nous devons reconnaître quelque vertu à ce projet de loi. Il s'agit d'un texte d'amélioration des conditions d'exercice du mandat local, d'un texte correctif, à défaut d'être structurant. Il ne créera pas des vocations d'élu par milliers,

Je pense aussi à l'introduction de la parité dans les fonctions exécutives pour les communes de plus de 1 000 habitants et aux progrès introduits en matière de représentation des femmes dans l'exécutif du conseil communautaire.

Concernant les pouvoirs de police du maire, nous sommes entrés dans le débat sans préjugés. Nous doutons qu'il faille donner toujours plus de responsabilités aux maires sans que les moyens soient au rendez-vous.

le compte rendu de l'action de la police et de la gendarmerie une fois par an devant le conseil municipal sera utile. Nous avons rassuré les acteurs associatifs en excluant les personnes sans domicile fixe du champ des amendes pour occupation illégale de la voie ou du domaine public.

des territoires plus ruraux, nous avons donné aux élus locaux un pouvoir d'initiative en matière de révision du schéma départemental de coopération intercommunale par le biais de la En ce qui concerne les droits des élus et la démocratie locale, nous avons obtenu que tous les adjoints puissent bénéficier des dispositions du code du travail pour ce qui est du droit à la suspension de leur contrat de travail et du droit à réintégration à l'issue de leur mandat. Nous avons obtenu que les conseillers communautaires en situation de handicap puissent se faire rembourser les frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique engagés pour l'exercice de leur mandat. Toutes ces avancées, l'adoption d'amendements de notre groupe, nous ont convaincus d'apporter notre appui au projet de loi ainsi modifié par le Sénat. Nous conservons cependant quelques regrets. Ainsi en est-il de la fin de la participation citoyenne dans les territoires. les dispositifs existants n'avaient pas empêché la crise des « gilets jaunes », mais leur suppression n'améliorera sans doute pas la situation. Des progrès supplémentaires auraient également pu être faits en matière de parité, avec le soutien de nombreuses associations d'élus et du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Le débat sur ce sujet reprendra sans doute à l'Assemblée nationale. Je veux aussi signaler que certains allers-retours en matière de dates ou de transferts de compétences pourraient créer quelques difficultés à l'avenir. Nous sommes trop nombreux, à droite comme à gauche, à regretter régulièrement l'instabilité de la loi pour nous satisfaire de changements de pied incessants. La si décriée loi NOTRe n'était certes pas parfaite, mais elle avait finalement été votée par presque tout le monde. Elle n'avait été repoussée que par quelques-uns ! Nous ! Il ne faudrait pas que les pommades inventées aujourd'hui pour soulager quelques irritations provoquent de nouvelles démangeaisons dans nos territoires

au département ou à la région des compétences qui leur ont été transférées par les communes. Alors que nos débats ont largement tourné autour du rôle central de la commune, vous avouerez, mes chers collègues, que la possibilité de transférer des compétences du bloc communal au département ou à la région sans l'aval des communes semble pour le moins discutable le moins discutable ... Les bonnes intentions concernant la rémunération des élus méritaient d'être étayées par des preuves d'amour supplémentaires. Nous sommes heureux pour les élus locaux que le Sénat se soit accordé sur une revalorisation du barème mieux adaptée aux capacités financières des communes de moins de 1 000 habitants,

avec plus de 1 900 conseillers régionaux, 4 000 conseillers départementaux et plus de 500 000 conseillers municipaux, la France est riche de 600 000 élus locaux, qui incarnent tous ses territoires. Les plus cyniques préfèrent mettre en avant le coût de ces élus pour les contribuables, sans mentionner le temps et le dévouement nécessaires pour assurer une fonction qui devient de plus en plus difficile. Je sais que je m'adresse, dans cette enceinte, à des convaincus, mais il fallait rappeler cette réalité, trop souvent occultée, caricaturée ou ignorée des grands médias. Certes, le présent projet de loi ne résoudra pas tout. Néanmoins, ne cachons pas la satisfaction que nous inspirent quelques avancées qui viendront faciliter le quotidien de nos élus. Je tiens, à ce titre, à saluer chaleureusement le travail de nos rapporteurs, Françoise Gatel et Mathieu Darnaud. Oui, les charges pesant sur les élus locaux n'ont cessé de s'alourdir ces dernières années, quelle que soit la majorité en place : baisse des dotations, transferts de charges, judiciarisation accrue Mais c'est sans doute la loi NOTRe qui cristallise le plus les mécontentements, en particulier s'agissant de la création forcée d'intercommunalités de taille disproportionnée. Certes, les maires ont su s'adapter aux regroupements et à la nouvelle répartition des compétences. Toutefois, ils ont avant tout besoin qu'on leur fasse confiance. Le maire doit retrouver sa place, au coeur de sa commune, naturellement, mais aussi, à l'avenir, au coeur de l'intercommunalité, quel que soit le poids de sa commune À cet égard, la conférence des maires, dont notre groupe défend l'instauration depuis longtemps, est, selon nous, le meilleur outil pour enrayer le sentiment légitime de dépossession éprouvé par de trop nombreux élus. sa création obligatoire, nous permettons à ces derniers d'être davantage informés sur les questions qui concernent leur territoire. Toutefois, nous le savons, pour que les plus petites communes renouent des liens de confiance avec l'intercommunalité, il est indispensable qu'elles y soient mieux représentées. égard, si le barème issu de la proposition de loi relative à la représentation des petites communes au sein des EPCI n'a pas été retenu, l'intégration de l'accord local est, quant à elle, bienvenue. Par ailleurs, il est heureux que nos débats aient montré qu'une intercommunalité apaisée est une intercommunalité qui n'agit que lorsqu'elle représente l'échelon le plus Cette logique de subsidiarité avait été oubliée, tout comme la réalité des territoires et de chaque commune. De ce point de vue, l'article 17, qui autorise le transfert de compétences entre collectivités, constitue, à nos yeux, une réponse adaptée. Par exemple, pour avoir sa propre géographie, l'eau implique une gestion qui ne correspond pas du tout aux frontières administratives. La suppression du transfert obligatoire de la compétence en matière d'eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, que notre groupe a soutenue, s'insère dans cette réalité d'une gestion différenciée des territoires qui va, finalement, dans le sens de l'histoire. Il en est de même des plans En commission, grâce à la sagesse des rapporteurs, nous avions voté un abaissement du seuil minimal de population des EPCI « XXL » afin de permettre à un plus grand nombre d'entre eux de créer des PLUI différenciés. séance plénière, le Sénat soit allé plus loin, en accordant davantage de latitude aux maires en matière d'urbanisme, que ce soit en instaurant à leur profit la possibilité de prendre l'initiative d'une modification simplifiée du PLUI si cette modification

deux catégories d'élus locaux coexistent, avec, d'un côté, des élus urbains, issus de communes largement dotées pouvant prendre en charge des dépenses comme celles de formation ou de déplacements et indemniser correctement leurs élus, et, de l'autre, des élus de communes rurales, faiblement dotées, qui, par souci de ne pas peser sur un budget limité, préfèrent ne pas demander la prise en charge de ces dépenses par leur commune. Telle est la réalité dans beaucoup de nos régions, ainsi que nos débats l'ont bien montré. Tout ne sera sans doute pas résolu dès le prochain renouvellement des conseils municipaux- ce n'est d'ailleurs pas la prétention des promoteurs de ce projet de loi -, mais des avancées notables ont vu le jour. les conditions indemnitaires des élus, je me réjouis que nous ayons permis une revalorisation à la fois adaptée, progressive et soutenable pour les plus petites communes.

Recueillent encore l'approbation des membres de mon groupe toutes les mesures visant à permettre aux élus de mieux concilier l'exercice de leur mandat avec leur vie familiale et professionnelle. Je pense, par exemple, à l'ouverture à leur profit du système de l'équivalence universitaire, que nous avons Nos débats sur la parité hommes-femmes ont également permis d'aboutir à des compromis qui viendront assurer une meilleure représentativité de nos conseils, en particulier en garantissant la parité pour les adjoints dans les communes de plus de 1 000 habitants. Enfin, quand les maires, jusqu'à présent à portée d'engueulade, deviennent à portée de bousculade, nous devons agir pour garantir leur protection. était-il d'important d'intégrer à ce projet de loi les dispositions législatives du plan d'action pour une plus grande sécurité des maires proposé par le président de la commission des lois. Les membres du groupe RDSE ont pris une part active à ces débats, en particulier nos chefs de file Nathalie Delattre et Henri Cabanel, que nous remercions. Nous nous félicitons de l'adoption de nombre de leurs amendements. À l'Assemblée nationale, désormais, de prendre ses responsabilités ! Pour l'heure, notre groupe votera ce texte, à une abstention près. La parole

le Sénat n'a été davantage le Sénat ! Deux semaines durant, dans cette enceinte, notre République décentralisée a subi un véritable contrôle technique. Deux semaines durant, nous avons évoqué la « sécabilité » des compétences déléguées, la problématique des périmètres intercommunaux ou encore la définition de l'intérêt communautaire : autant de questions dont l'examen est la raison d'être de notre assemblée,

De ce tohu-bohu législatif, que reteindront nos concitoyens, mes chers collègues ? Après tout, l'intercommunalité n'est pas leur langage, non plus que le coefficient d'intégration fiscale ou la compétence relative à la promotion du tourisme

les complications et les mésaventures de la décentralisation, mais le fond de notre affaire doit rester les Français. Monsieur le ministre, vous avez remis l'ouvrage sur le métier. Vous nous invitez même à légiférer sur le montant des indemnités de fonction. C'est dire si vous aimez vivre dangereusement Avec ce texte, vous souhaitez assurer le service après-vente de la loi NOTRe, mais pas de n'importe quelle manière. Des règles du jeu ont été fixées : oui à des assouplissements correctifs, non à un nouveau big-bang territorial aux accents wagnériens. Au fond, je déduis de votre projet de loi trois impératifs : libérer, protéger, simplifier. D'abord, ce texte vise à libérer, mais pas au nom de n'importe quelle liberté,

Nous ne décentralisons pas aujourd'hui qu'avec des décentralisateurs ! J'en veux pour preuve quelques opérations clandestines- je pense à l'amendement relatif à la police municipale à Paris voire folkloriques, allant de l'abrogation de la loi NOTRe à l'abaissement du droit de vote à 16 ans, qui, sur un malentendu, n'étaient pas loin de « glyphosater » le texte. La liberté, c'est davantage l'assouplissement des conditions de délégation de compétences entre collectivités ou encore la faculté, pour les départements, d'attribuer des aides aux entreprises. ce texte vise à protéger. L'élu local exerce une profession risquée. Nous devons lui prêter main-forte et le remercier. À ce titre, les pouvoirs de police du maire ont été renforcés. L'autorité du maire, officier de police judiciaire, a été restaurée. L'engagement des élus a été mieux reconnu. La conciliation entre le mandat local et la vie professionnelle a été favorisée.

d'administrer un choc de simplification pour desserrer le garrot normatif qui polytraumatise nos élus. De grâce, cessons d'appeler « vides juridiques » leurs espaces de liberté

la période des vendanges est désormais terminée. Je veux dire aux maires que je veillerai à ce que ce texte prépare, avec un peu de réussite, la République de demain. Monsieur le

si vous disposez d'une délégation de vote, le nom du sénateur pour lequel vous devez voter s'affiche automatiquement sur le terminal de vote au-dessous de votre nom. Vous pouvez alors voter pour vous-même et pour le délégant en sélectionnant le nom correspondant, puis en choisissant une position de vote. Si vous avez donné une délégation et que vous êtes finalement présent, vous pouvez voter directement en insérant votre carte dans votre terminal de vote. La position de vote alors exprimée primera sur un vote exprimé par délégation.

deux objectifs majeurs au titre de l'examen des quelque 1 000 amendements. Premièrement, il convenait d'éviter de reproduire les errements de la loi NOTRe en créant des sources de déstabilisation majeure pour le prochain mandat municipal. Une génération d'élus, entre 2014 et 2020, aura déjà connu beaucoup de modifications institutionnelles. Il ne s'agissait pas de réserver à la génération 2020-2026 la même instabilité et les mêmes écueils. Deuxièmement, il importait de connecter les questions institutionnelles et juridiques aux questions financières.

invite à l'engagement résolu de la France en faveur de toute initiative concertée au niveau européen et international de nature à faire cesser l'offensive menée par la Turquie au nord-est de la Syrie.

kurdes, nouvelles Antigone de la résistance, de la dissidence. Enfin il y eut Raqqa. Si les forces démocratiques syriennes à majorité kurde

moralement injustifiable, parce qu'il s'agit, ni plus ni moins, d'un nettoyage ethnique, avec son cortège d'horreurs, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité.

Mes chers collègues, cette proposition de résolution vise à affirmer solennellement que nous n'oublions pas les Kurdes qui ont payé le prix du sang pour nous, Européens et Français.

Pour l'avenir, je fais trois propositions. La première concerne la coalition : le moment est venu pour elle d'actualiser sa stratégie. Où voulons-nous aller ? Par quels moyens voulons-nous poursuivre

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de résolution qui nous est soumise invite à l'engagement résolu de la France en faveur de toute initiative concertée au niveau européen et international de nature à faire cesser l'offensive menée par la Turquie au nord-est de la Syrie. Nous ne pouvons bien évidemment que souscrire à cette pétition de principe et renouveler, à cette occasion, la condamnation la plus totale de l'agression criminelle de la Turquie, rendue possible par le « feu vert » américain de Donald Trump. Mais, nous l'avons dit dès le premier jour, les pétitions de principe, les condamnations verbales ne suffiront pas à arrêter le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. À quelques heures maintenant de la fin d'un cessez-le-feu précaire qui peut signifier la reprise d'un massacre à grande échelle des Kurdes et des populations et des réfugiés du nord-est de la Syrie, notre inquiétude est à son comble. Erdogan vient, semble-t-il, de rejeter la proposition de prolongation du cessez-le-feu faite par le Président de la République Emmanuel Macron à Vladimir Poutine. La pression ne doit donc pas se relâcher, mais s'amplifier encore pour éviter le pire. Plus que jamais, tout doit être fait pour sauver nos amis Kurdes et les populations installées ou réfugiées dans le nord-est de la Syrie. Si les mots ont un sens,

La France n'est pas à la hauteur du péril. Tout se passe en effet comme si, derrière les mots de condamnation, nous étions en train de lâchement abandonner les Kurdes et les forces démocratiques syriennes. Ces forces combattantes et les populations civiles sont à la merci du feu de l'armée et des bombardiers turcs. Erdogan veut liquider physiquement l'expérience du Rojava démocratique- dont le compte twitter est actuellement bizarrement bloqué

Où sont les sanctions économiques et politiques fortes contre le régime d'Ankara que nous réclamons depuis le premier jour ? Erdogan a aussi redoublé, ces derniers jours, la répression contre les Kurdes en territoire turc. Devant ces nouvelles alarmantes et concordantes, qu'a annoncé Emmanuel Macron au Conseil européen ? Une possible rencontre à Londres entre Boris Johnson, Angela Merkel, lui-même et Erdogan, mais pour quoi faire ? Pour colmater les brèches et reconstituer une coalition avec celui-là même qui massacre les Kurdes et les forces démocratiques syriennes ? Ces hypocrisies doivent cesser Nous restons enlisés dans l'OTAN, avec des alliés qui nous ont tourné le dos, et nous perdons un temps précieux pour parler à nouveau d'une voix indépendante dans le monde, pour mobiliser l'ONU et retrouver une crédibilité mise à mal par ce qui vient de se passer L'« engagement résolu de la France », ce devrait être aussi un soutien sans faille aux acteurs humanitaires et aux principes que quinze ONG ont rendus publics la semaine dernière, notamment pour garantir l'accès sans entrave des secours humanitaires à toutes les zones du conflit. Les bombardements turcs occasionnent de nouveaux dégâts insupportables. L'utilisation d'armes explosives dans les zones peuplées continue ; nous ne pouvons l'accepter. En avançant, les forces turques risquent de priver de toute aide humanitaire des centaines de milliers de personnes supplémentaires, mettant leur vie en péril, ou de les conduire à prendre de nouveau la route de l'exil. Mais vers où ? Vers quel nouvel enfer ? La France doit agir sans tarder aux côtés de ces ONG pour obtenir ce qu'elles demandent. Enfin, j'aborderai une question que je sais plus difficile

ne pas dire plus, devant la démarche entreprise par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en Irak. Sous prétexte de les maintenir en sécurité, nous tentons, semble-t-il, de sous-traiter le gardiennage de ces Les conditions de ce marchandage semblent peu reluisantes. Est-ce responsable, est-ce digne de la France ? Je pose la question. Le coordonnateur des juges antiterroristes, David de Pas, vient, tout à fait exceptionnellement, de s'en inquiéter publiquement et plaide pour le rapatriement des djihadistes français. Selon lui, « la question du rapatriement est un enjeu de sécurité et de justice à long terme ».

Pourquoi s'obstiner à refuser leur rapatriement alors que celui est demandé par l'ONU, par la Commission nationale consultative des droits de l'homme et par les ONG travaillant sur cette question, au nom de toutes les conventions internationales protégeant les droits de l'enfant dont nous sommes signataires ? Qu'attendons-nous ? Leur mort lente ou leur retour dans les griffes de Daech ? Ce sont des questions difficiles, mais il faut avoir le courage de les poser

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la Turquie a lancé, le 9 octobre dernier, l'opération « Source de paix un paradoxe ! -dans le Kurdistan syrien. Ankara dit vouloir protéger sa frontière contre les terroristes. Pourquoi un pays ami, membre de la coalition internationale contre Daech, également membre de l'OTAN, engage-t-il un conflit armé de manière unilatérale, sans le moindre accord officiel avec ses alliés ? Les motifs de l'opération ne sont peut-être pas encore totalement connus. Ces dernières années, nous avons vu le comportement d'Ankara changer. Alors que le pays est membre de l'OTAN et candidat à l'adhésion à l'Union européenne, son dirigeant a tenu hier Tout l'Occident s'est rangé aux côtés des terroristes et ils nous ont attaqués tous ensemble. Parmi eux les pays de l'OTAN, les pays de l'Union européenne. Tous. » Ce n'est pas parce qu'un djihadiste est français que tous les Français sont des terroristes : il en est de même pour les Kurdes ! Cette incursion dans une région kurde de Syrie risque de tourner au massacre. Une enquête de l'Office pour l'interdiction des armes chimiques a été ouverte vendredi dernier : du phosphore blanc aurait été utilisé contre les Kurdes. Cette offensive est injustifiable parce qu'elle a lieu contre des alliés dans la lutte contre Daech. Les Occidentaux ont déployé des forces aériennes et des unités des forces spéciales, dont nous saluons l'engagement et le courage. Les Kurdes, soutenus par nos soldats, se sont courageusement battus contre Daech et ont largement contribué à sa défaite territoriale. Bien sûr, les Kurdes se sont battus pour leur survie, comme l'a cyniquement rappelé le président Trump. Ils se sont battus aussi pour la survie de ceux qu'ils auraient pu abandonner, comme d'autres l'ont fait. Lorsque, en 2014, 50 000 Yézidis se sont trouvés piégés sur le mont Sinjar -plusieurs milliers d'entre eux furent massacrés ou convertis de force et réduits à l'esclavage par les djihadistes -, ce sont les forces kurdes qui ont permis leur évacuation. Les Kurdes se sont battus pour leur survie, certes, mais nous savons aussi ce que la sécurité de notre pays doit à leur engagement. Cette offensive est injustifiable parce qu'elle vise ceux que la Turquie a déjà abandonnés sous les coups des djihadistes. Il faut se rappeler que, à la fin de l'année 2014, Daech assiégeait la ville kurde de Kobané, qui se trouve à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Durant le premier mois, la Turquie, pourtant membre de la coalition internationale engagée dans la lutte contre Daech, n'avait pas réagi. Pis, elle avait fermé sa frontière et empêché les forces kurdes de recevoir des secours, des renforts et des armes. À cette époque déjà, la Turquie avait tenté d'obtenir, en échange de l'ouverture de sa frontière, la création d'une zone tampon large de vingt kilomètres le long de sa frontière syrienne.

nombreux acteurs y sont présents. La solution ne pourra être que politique. Le principe de l'intangibilité des frontières n'est pas absurde, mais celui de l'autodétermination des peuples non plus. Le Kurdistan, c'est de 40 millions à 50 millions de personnes réparties entre quatre pays. Pour rappel, la Syrie compte 20 millions d'habitants et l'Irak 40 millions. Contre le régime de Saddam Hussein en 2003, contre Daech au Levant et, n'en déplaise aux propagateurs de, y compris durant la Seconde Guerre mondiale, les Kurdes ont maintes fois prouvé qu'ils étaient des alliés efficaces, fiables et loyaux. Nous ne souhaitons pas voir la Turquie s'éloigner de ses alliés. De même, nous ne souhaitons pas voir les États-Unis s'éloigner des leurs. La volte-face américaine est très surprenante. C'est un déchirement pour les militaires de lâcher les troupes kurdes aux côtés desquelles elles ont combattu. Le retrait américain entraîne celui des Occidentaux, faute de moyens. Voilà encore la preuve qu'il est urgent, pour l'Europe, d'atteindre l'autonomie stratégique. L'Union européenne prend conscience qu'elle doit affronter cette situation sans l'appui des États-Unis, puisque Donald Trump poursuit la stratégie, engagée sous Barack Obama, de désengagement américain du Moyen-Orient. L'Union européenne est aujourd'hui confrontée aux conséquences de ses erreurs, au premier rang desquelles la sous-traitance. Faute de trouver une solution pour ses ressortissants djihadistes, elle a sous-traité leur traitement judiciaire, devenant ainsi l'otage de ceux qui les détiennent et qui peuvent faire du chantage à leur libération ou à leur expulsion. C'est une erreur que ni les Russes ni les Américains n'ont commise, puisqu'ils ont, eux, rapatrié leurs ressortissants djihadistes. Pour ne pas avoir à gérer elle-même ses frontières, l'Union européenne a sous-traité le contrôle des réfugiés à la Turquie. Ankara fait logiquement du chantage pour obtenir ce qu'elle veut de l'Europe. L'Europe, par absence de courage et de volonté politique, se retrouve maintenant otage d'acteurs qui ont assumé pour elle une part de ses responsabilités. Ce n'est pas la première fois que les Européens se condamnent à l'impuissance. Lors de la crise géorgienne, de celle de l'Ukraine, des attaques chimiques en Syrie, à propos de l'accord sur le nucléaire iranien, l'Europe n'a pas su montrer sa puissance. La cause en est toujours la même : la désunion. La crise actuelle ne fait pas exception, les Européens sont profondément divisés, la Hongrie ayant ainsi apporté son soutien à Erdogan. Ce n'est pas la première fois non plus que les Kurdes sont abandonnés à leur sort. La revue stratégique avait mis en évidence l'instabilité et l'insécurité qui caractérisent notre XXIsiècle. Nous y sommes, et ce dans bien des domaines Le président Erdogan a annoncé aujourd'hui que l'offensive reprendra « avec une plus grande détermination » faute d'un retrait kurde. Ce chantage est totalement inadmissible.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, malgré nos alertes et celles de nos alliés, des militaires turcs et leurs supplétifs syriens ont pénétré, mercredi 9 octobre dernier, dans le nord-est de la Syrie dans le cadre d'une offensive lancée par Ankara pour, officiellement, se protéger des « terroristes » kurdes. Dimanche, soit trois jours avant l'offensive, le président Trump avait annoncé, sans nous en avertir au préalable, le retrait immédiat de ses troupes de Syrie, alors que les Américains sont les alliés, sur place, des forces démocratiques syriennes, composées majoritairement de Kurdes, mais également d'Arabes et de chrétiens, dans la lutte contre Daech. C'est bien leur départ qui a permis l'offensive turque, avec les conséquences humanitaires, politiques et stratégiques que l'on connaît. Cet acte est une faute morale à l'égard de nos alliés des forces démocratiques syriennes, qui ont payé le prix fort de la lutte contre Daech sur le terrain. Sans eux, l'État islamique n'aurait pu être vaincu militairement comme il l'a été. C'est également une faute politique et stratégique.

L'Union européenne a exigé l'arrêt de l'offensive et le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence, le 10 octobre, mais sans résultat concret.

Ce nouvel épisode du conflit syrien est en outre lourd de conséquences pour l'équilibre global des puissances. En effet, l'attaque par la Turquie de forces alliées aux Américains et soutenues par une coalition occidentale n'a pas manqué de jeter le trouble dans l'Alliance atlantique, dont sont membres à la fois Washington, Ankara et nous autres européens. Elle met donc dangereusement en évidence les failles du camp occidental. Que valent aujourd'hui

En effet, les forces kurdes, lâchées par leurs alliés américains et auxquelles le soutien de la coalition ne peut suffire, ont été contraintes de conclure un accord avec leurs ennemies d'hier, les forces du régime de Bachar el-Assad,

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'invasion par la Turquie du nord-est de la Syrie, sur une bande

lorsqu'ils ont pris, pour le premier, et cautionné, pour le second, cette décision catastrophique. Pourtant, les conséquences en seront internationales et géopolitiques. Elles s'étendront sur le court, le moyen et le long terme. Les conséquences de court terme sont connues, elles ont été largement présentées, avec émotion, par le président Retailleau. Il s'agit, bien sûr, de la trahison par les États-Unis de nos alliés kurdes, dont les efforts ont été si précieux pour réduire le califat territorial de Daech. Il s'agit aussi de la remise en selle de Daech, qui n'en espérait sûrement pas tant des Occidentaux ... Sur le moyen terme, ces événements marquent un tournant majeur pour trois raisons. Ils marquent tout d'abord la victoire du régime de Bachar el-Assad et de ses soutiens iranien et russe. C'est la fin du processus de Genève et de l'espoir d'une solution politique à la guerre civile syrienne. à la guerre civile syrienne. Ils symbolisent ensuite le désengagement américain du Moyen-Orient et leur refus d'assumer la responsabilité de la sécurité collective dans cette région ô combien stratégique du monde. Les Américains abandonnent ce rôle à la Russie, ce qui n'a échappé à personne dans la région. Pour dire les choses simplement, les Américains ont livré le Moyen-Orient sur un plateau aux présidents Poutine et Rohani.

En faisant le jeu russe, en attaquant nos alliés kurdes, en permettant la résurgence de Daech et en nous menaçant d'un chantage aux réfugiés, la Turquie est entrée dans l'isolement. Après la remise en cause des libertés publiques, après l'achat des systèmes de défense antiaérienne S400 à la Russie, après les forages illégaux au large de Chypre, la Turquie achève de tourner le dos à l'Europe. Là encore, les conséquences seront très lourdes Enfin, il y a les conséquences de long terme. Cette crise est le fruit du « pivot stratégique » vers l'Asie organisé par les Américains, annoncé par Barack Obama et accéléré par Donald Trump l'Europe et le Moyen-Orient ne sont plus des priorités stratégiques pour les États-Unis. Ce retrait américain laisse apparaître l'Europe dans toute sa faiblesse stratégique et pose une forte question à l'OTAN. Aujourd'hui, l'OTAN n'a aucune autonomie par rapport aux États-Unis, comme l'a illustré l'indigence des réponses que son secrétaire général, M. Stoltenberg, avait à présenter lorsque je l'ai moi-même interpellé à Londres sur ce sujet il y a une semaine. Pourtant, à part les États-Unis et la Turquie, l'ensemble des alliés condamnaient cette attaque. Pouvons-nous agir sans les Américains ? Je souhaite que ces événements, qui inquiètent tous les pays européens,

L'enjeu, pour les Européens, est de construire ensemble leur sécurité. Nous commençons à peine à partager l'analyse des menaces. Pendant longtemps, on opposait deux Europe : une Europe de l'Ouest, préoccupée surtout de la menace au Sud, et une Europe de l'Est, préoccupée surtout par l'action déstabilisatrice de la Russie. la Russie. Nous constatons tous que cette opposition n'a plus lieu d'être. L'acteur principal aujourd'hui en Syrie, celui devant qui les États-Unis ont choisi de s'effacer, c'est la Russie. Ce qui se passe en Syrie a des conséquences pour l'Europe, tout comme ce qui se passe en Irak, au Sahel, en Ukraine ou en Géorgie. C'est d'ailleurs pour cela qu'il convient de parler à la Russie Aujourd'hui, nous sommes encore très loin de pouvoir imaginer des opérations militaires européennes d'envergure, mais je ne doute pas que le drame kurde va accélérer le réveil stratégique de beaucoup d'Européens. Dans un monde où l'égoïsme et le court-termisme électoraliste deviennent les seuls axes de la politique étrangère, dans un monde où le jeu des puissances broie sans états d'âme le droit international, mais aussi, hélas, les populations civiles, ceux qui ne seront pas capables de se défendre par eux-mêmes s'exposeront à être délaissés, abandonnés, trahis et enfin soumis. Nous le disons solennellement : il s'agit, pour l'Europe, de ne pas sortir de l'histoire. Oui, mes chers collègues, les auteurs de la proposition de résolution ont raison d'affirmer que la France doit s'engager résolument pour les Kurdes. Tout l'y conduit : l'honneur, d'abord, qui fait que l'on n'abandonne pas ses frères d'armes ; notre sécurité à court terme, ensuite, puisqu'il s'agit de freiner, voire d'empêcher, si c'est possible, le retour de Daech notre sécurité sur le long terme, enfin, car il faut sans plus attendre travailler d'arrache-pied avec nos amis Européens pour redéfinir notre architecture de sécurité collective. Quel rôle pour l'OTAN, qui a pour l'instant surtout montré ses limites ? Quelles capacités militaires pour les Européens ? Quelle autonomie stratégique, à un moment où nous voyons qu'il faut d'abord compter sur nous-mêmes ? Ce sont toutes ces questions que pose la tragédie des Kurdes. La proposition de résolution qui nous est présentée est un jalon sur une route qui sera longue. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera naturellement la proposition de résolution et travaillera, dans les mois qui viennent, avec tous ceux qui, au Sénat, partagent le sentiment de l'urgence du réveil stratégique. Je salue le consensus politique très large que cette proposition de résolution a fait naître au Sénat. Aujourd'hui, mes chers collègues, nous parlons d'une voix forte, unie, parce que défendre les Kurdes, c'est défendre notre honneur, parce que défendre les intérêts de la France, c'est aussi agir pour la sécurité des Français

Il existe des événements glorieux, et d'autres qui parfois le sont moins. Il existe des moments sur lesquels les nations se retournent avec regret, trop longtemps après. Mais les moments où un simple choix peut faire basculer dans l'honneur ou le déshonneur sont rares. Notre pays est aujourd'hui devant l'un de ces moments, au regard de l'offensive turque dans le nord-est syrien, qui expose en première ligne le peuple kurde. Depuis 2011, la Syrie est en guerre civile. Dans l'intervalle, notre pays, comme d'autres, a été durement touché par le terrorisme de Daech. Dès 2013, avant les volte-face américaines avaient empêché la communauté internationale de se prémunir contre les crimes d'Assad et le développement de l'État islamique. Nous connaissons tous cette histoire.

: fermer les yeux, c'est laisser déstabiliser la région, c'est permettre aux cellules toujours actives de Daech de se restructurer, c'est mettre à mal la sécurité de nos concitoyens ; fermer les yeux, c'est abandonner les Kurdes, c'est trahir un allié alors qu'on a déjà vu le sort réservé aux Kurdes à Afrin, il y a un an et demi ; fermer les yeux, c'est redonner la main à Assad, c'est lui pardonner ses crimes contre son propre peuple ! Si les États-Unis ont une responsabilité évidente, ne rien faire serait, pour la France, particulièrement déshonorant.

alors eu les honneurs de la communauté internationale, comme en 2004, avec le refus de Jacques Chirac d'engager la France dans une guerre dangereuse et sans fondement. Il est temps que notre pays agisse ! C'est ce que propose cette résolution. Le Gouvernement de la France doit tenir compte de cette résolution et agir enfin, même si c'est avec retard. J'irai même plus loin, monsieur le secrétaire

Notre pays doit demander à l'Union européenne des sanctions fortes à l'encontre de la Turquie, à l'image de ce qui avait été fait contre la Russie. Notre pays doit promouvoir une initiative devant l'ONU pour que la zone tampon soit rétablie et contrôlée par des forces internationales. Notre pays doit agir auprès de l'OTAN face à cette attaque de la Turquie contre un de nos alliés dans la guerre contre Daech. L'urgence est réelle. Les combats ont déjà fait des centaines de morts et déplacé 300 000 personnes, qui s'ajoutent aux 3,6 millions de réfugiés syriens que la Turquie a accueillis sur son territoire. La situation sera bientôt inextricable si nous n'agissons pas rapidement. Mes chers collègues, je conclurai par un mot sur la situation internationale, bien au-delà de celle du peuple kurde, qui nous préoccupe grandement. À force d'intérioriser une certaine forme d'impuissance, la France, l'Europe, nos alliés, plus personne n'agit lorsqu'un conflit s'ouvre quelque part dans le monde. La communauté internationale est devenue passive,

devons réagir. Ce mutisme croissant devant les violations du droit international, cette lente agonie de résolutions inappliquées face aux conflits locaux n'apportent rien de bon pour la paix et l'équilibre mondial.

monsieur le secrétaire d'État, je le prononce avec regret. Mais est-il possible, aujourd'hui, d'en employer un autre, alors que la France et l'Union européenne en sont réduites au rôle de spectateurs passifs d'un nouveau drame dans un territoire ensanglanté par la guerre civile depuis 2011 ? L'intervention de l'armée turque dans le nord-est de la Syrie, facilitée par le feu vert du président des États-Unis, permet à Vladimir Poutine d'apparaître désormais comme le maître du jeu dans un conflit ô combien complexe, dont chacun mesure les effets dévastateurs. Sur le plan humanitaire, tout d'abord : une fois de plus, nous voyons des populations civiles ballotées, déplacées, menacées. La progression rapide des forces turques aurait déjà conduit au déplacement de 130 000 personnes, et je préfère ne pas compter le nombre des morts d'un bilan provisoire, compte tenu de l'implication, aux côtés des forces loyalistes, de milices supplétives animées par une soif sanguinaire de vengeance. Nous gardons tous à l'esprit les massacres de civils, de Yézidis ou de membres de tribus sunnites hostiles à Daech notamment, le commerce des femmes, les pillages, les déplacements forcés de populations, et autres violences commises au nom d'un obscurantisme mortifère que Daech a porté à son paroxysme. En nommant cette organisation, qui mène contre l'Occident et ses valeurs une guerre sans merci, aveugle et sauvage, j'aborde un deuxième effet de l'inconséquence de Trump et d'Erdogan. Certes, ce dernier s'est dit « prêt à écraser les têtes des terroristes », mais sa déclaration, mes chers collègues, vise principalement les Kurdes, nos alliés, avec lesquels nous avons gagné une bataille contre l'État islamique

En visant l'administration autonome installée dans le nord-est de la Syrie, qu'il considère comme une base arrière du Parti des travailleurs fragilisé par la situation économique de son pays et par les résultats des récentes élections municipales, a choisi la fuite en avant. nous avons un devoir moral envers nos frères d'armes kurdes. Les combattants et les combattantes des forces démocratiques syriennes ont permis, avec les forces de la coalition internationale, de détruire la tentative d'organisation territoriale des fanatiques islamistes de Daech. Cette calamiteuse opération turque soulève également des enjeux sécuritaires ; ses effets sont substantiels pour le Proche-Orient et le Moyen-Orient, mais aussi du point de vue de nos propres intérêts. Le Premier ministre l'a rappelé ici même, mercredi dernier, en évoquant clairement le risque d'une résurgence des effectifs et des forces de Daech. cette zone se trouvent 10 000 djihadistes et près de 2 000 prisonniers contrôlés par les forces démocratiques syriennes. Nous avons laissé dans la région de bien encombrants détenus djihadistes français que nous souhaiterions voir juger en Irak. est la position de la France, monsieur le secrétaire d'État, et le RDSE la partage. Il nous faut des garanties, d'une part, quant à la capacité de l'Irak à juger sur place les crimes commis par les détenus français, et, d'autre part, sur les conditions de leur confinement, afin d'éviter leur évasion, rendue possible dans le contexte actuel. Il semblerait que des familles de djihadistes aient pu s'échapper, notamment du camp d'Ayn Issa. Combien

réfugiés. Cet enjeu ne concerne pas seulement la Turquie : le président Erdogan nous le rappelle assez souvent, menaçant de nourrir davantage la crise migratoire européenne s'il n'obtenait pas plus de soutien sur ce volet. L'aide financière apportée par l'Union européenne ne semble pas suffire à calmer Ankara, qui voit dans son opération en Syrie le moyen de relocaliser Dois-je ici revenir sur les palinodies d'une Union européenne qui, une fois de plus, n'est pas parvenue à un accord sur la suspension des contrats d'armement avec la Turquie ? Une telle mesure serait pourtant, à ce stade, ô combien symbolique ! Quant aux sanctions économiques, évoquées par certains, elles affecteraient en premier lieu l'Allemagne et la France. Je me répète donc, mes chers collègues : chaos, impuissance, colère. Cela dit, devons-nous baisser les bras, nous lamenter et laisser la fragmentation, les menaces et la brutalité l'emporter sur la diplomatie et la raison ? Évidemment non

Nous avons très certainement péché de n'avoir pas porté avec suffisamment de courage et d'audace les propositions politiques indispensables à la sortie des conflits. jusqu'aux élections de novembre 2020, les Américains se retireront des zones d'intervention pour mieux se recroqueviller sur leurs problèmes intérieurs.

si- je l'accorde -notre attachement au respect des droits de l'homme nous impose des contraintes bien légitimes. Aux maux de l'asservissement et de la tyrannie, opposons démocratie, courage, responsabilité et, malgré tout, espoir.

je tiens à saluer l'inscription à l'ordre du jour de nos travaux de ce débat sur un dossier tragique. Il nous permet de nous prononcer sur l'offensive massive et sanglante menée par la Turquie et ses supplétifs dans le nord-est de la Syrie contre les combattants kurdes. Notre émotion est vive,

Notre groupe condamne avec fermeté et gravité cette opération militaire lancée par la Turquie depuis quatorze jours ; cette violation flagrante du droit international doit cesser.

parce que cette offensive a été lancée contre des femmes et des hommes qui sont nos alliés dans la lutte contre le terrorisme, au sein de la coalition internationale mise en place par les États-Unis en 2014 et dont la Turquie fait partie.

Sans leur aide décisive et sans leur sacrifice ultime, nous n'aurions pu aboutir aussi vite à la fin de la bataille territoriale contre Daech en Syrie et à la libération de l'Irak.

quelle confiance et quelle crédibilité peut-on accorder à une alliance militaire si elle débouche inopinément sur une telle trahison ?

Le risque de résurgence de Daech sur les cendres de ce chaos est élevé, et la Turquie porte désormais une forte responsabilité. Comment parler de « grand jour pour la civilisation », comme l'a fait le président des États-Unis, au sujet d'une trêve négociée en l'absence des principaux acteurs concernés et entérinant une capitulation devant les revendications turques ? Avec l'inconstance du président Trump, qui s'est brusquement ravisé pour imposer un accord précaire, c'est la crédibilité occidentale, celle de l'Alliance atlantique et du monde libre face au totalitarisme, qui se trouve affaiblie.

Nous ne pouvons plus faire l'économie d'une autonomie stratégique européenne, telle que défendue par le Président de la République son agenda de renforcement de la souveraineté européenne. Notre groupe sait déjà pouvoir compter sur la détermination résolue du Gouvernement à s'engager « en faveur de toute initiative concertée au niveau européen ou international visant à mettre un terme à l'offensive militaire » turque. C'est pourquoi il soutiendra cette proposition de résolution. Nous devons multiplier les efforts diplomatiques, en étroite coordination avec nos partenaires de la coalition anti-Daech, dans le cadre de l'Union européenne, de l'OTAN et du Conseil de sécurité. La voie diplomatique est la seule qui doive être empruntée pour régler ce conflit. Le Président de la République a dernièrement annoncé une initiative commune avec la Chancelière allemande et le Premier ministre britannique en vue de rencontrer le président turc en marge du sommet de l'OTAN de décembre. Nous nous en félicitons et espérons qu'une démarche forte permettra d'avancer vers la résolution de ce conflit. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, si nous sommes devant une situation absolument inextricable au Moyen-Orient, ce n'est pas seulement la faute des pays concernés. C'est aussi et surtout la faute des pays occidentaux. Pourquoi l'État islamique est-il apparu et s'est-il développé ?

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le retrait brutal des forces américaines du nord de la Syrie, suivi du déclenchement des hostilités par la Turquie, est un nouveau tournant dans ce conflit vieux de plus de huit ans. La décision de retrait des Américains n'est pas une réelle surprise, puisqu'elle prolonge une volonté de désengagement déjà annoncée par le président Obama, que son successeur aura mise en à sa façon, avec brutalité et précipitation, mettant fin, par la même occasion, à une politique néoconservatrice américaine de plus de quinze ans au Moyen-Orient. Rarement une escalade politico-militaire aura provoqué autant d'effets collatéraux et fait surgir autant d'interrogations. C'est d'abord l'OTAN qui voit se confronter les positions de deux de ses principales composantes. Les interrogations sur cette institution, dont l'objet même est d'être une instance politico-militaire de sécurité collective, ne datent pas d'aujourd'hui, même si les critiques se devaient jusqu'à présent

Une deuxième question a trait bien évidemment à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'État syrien. Les conflits de Syrie et d'Irak auront montré l'importance cruciale de l'unité et de l'intégrité territoriale de ces pays.

Il est primordial que tout soit fait pour que le déclenchement des opérations turques visant à installer une zone de sécurité ne soit pas le prétexte à une remise en cause de l'intégrité territoriale de la Syrie.

Les discussions d'Oslo avaient laissé entrevoir une ouverture possible ; les événements de Kobané auront brutalement rappelé que, pour les Turcs, le PKK est le premier adversaire, bien avant Daech.

L'offensive engagée le 9 octobre dernier procède de la même logique : reprendre possession d'une bande frontalière pour y installer des réfugiés. Mais la réalité du terrain, selon les retours que nous en avons, donne peu de crédit à une telle affirmation. affirmation. Quand on sait le prix de l'engagement et du sang versé par les combattants kurdes dans la lutte contre Daech, la sécurité est la moindre des marques de reconnaissance qui leur sont dues. Les circonstances de la guerre, qui ne sont pas à l'honneur des Occidentaux, Français compris, auront conduit les Kurdes à trouver un accord avec les autorités syriennes. Cet accord ne leur offre pas pour autant les garanties nécessaires face aux opérations turques. Il est donc important que tout soit fait pour mettre un terme à l'engagement militaire turc sur le sol syrien, seule garantie pour l'avenir des populations, quelles que soient leurs composantes ethniques et religieuses. On ne saurait évoquer le nord de la Syrie sans parler des prisonniers, qui sont quelques dizaines de milliers, dont un nombre important d'Occidentaux et de Français. Les accords conclus entre les forces kurdes et les autorités syriennes prévoient de sécuriser les camps de prisonniers, dont on pourrait craindre la dispersion, avec toutes les conséquences que cela

au regard tant de considérations humanitaires que du risque de voir se développer une génération d'enfants soldats. C'est une question sensible, mais l'enjeu sécuritaire, au-delà de l'aspect humanitaire, impose la prise de décisions politiques courageuses. Dans ce conflit qui n'est pas encore terminé, et au sein duquel le combat contre Daech reste total, même s'il prend une forme nouvelle, l'Union européenne aura été, une fois de plus, la grande absente,

Féraud. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, chers collègues, la semaine dernière, nous sommes nombreux à avoir interpellé le Gouvernement sur la réponse que la France doit apporter à l'agression militaire turque. les troupes d'Erdogan ont envahi le nord de la Syrie, en complète violation du droit international et à la suite d'une nouvelle volte-face du président Trump, qui confine à la trahison. En visant les Kurdes du Rojava, qui ont combattu si courageusement et si efficacement à nos côtés, le président turc a mis à mal une situation déjà très fragile

N'oublions pas les crimes de guerre qui sont commis depuis quelques jours dans le nord de la Syrie ; n'oublions pas non plus que les supplétifs de l'armée turque sont des milices islamistes. Je veux remercier le président Retailleau d'avoir pris l'initiative de cette proposition de résolution, que j'ai cosignée avec Patrick Kanner et Christian Cambon. Elle vise à engager la France dans la recherche d'une sortie de cette situation dramatique, une situation profondément injuste quand on connaît l'engagement des Kurdes aux côtés de la coalition internationale contre Daech et particulièrement dangereuse pour l'avenir, tant elle nous affaiblit face au terrorisme islamiste. Certes, la situation géopolitique est complexe, et le nord-est syrien est aujourd'hui au carrefour de toutes les influences qui s'exercent au Moyen-Orient. Certes, les présidents américain et turc ont pris des décisions très néfastes, chacun pour des raisons de politique intérieure. Certes, l'Iran constitue sans faiblir un axe chiite, porteur, d'ailleurs, de graves conflits à venir. Certes, la Russie, quant à elle, poursuit avec détermination une politique cynique et brutale de soutien au régime syrien, en cohérence avec ses ambitions régionales, tandis que l'Europe reste faible de ses divisions et de son manque d'ambition.

choix. Le message que nous adressons ici, c'est celui du refus du fatalisme, car l'Europe n'est faible que de son manque de volonté. Aujourd'hui, seule la France peut, avec l'Allemagne, l'entraîner à affirmer la défense de ses valeurs, de ses alliés et de ses intérêts. Sanctions économiques contre un pays, la Turquie, largement dépendant de ses échanges avec l'Europe, sanctions contre les dirigeants turcs détenant des avoirs à l'étranger, demande de suspension de la participation de la Turquie à l'OTAN, arrêt des négociations d'adhésion à l'Union

Je rappellerai la résolution 688 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée en avril 1991, qui permit l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne dans le nord de l'Irak.

Or en attaquant les Kurdes, la Turquie nous a attaqués nous-mêmes, d'autant que nous leur sous-traitons la prise en charge des prisonniers djihadistes. Erdogan comprend très bien le langage de faiblesse. Nous devons sortir de la posture défensive et de l'impasse dans lesquelles nous nous sommes nous-mêmes placés. Cette proposition de résolution vise à encourager la France à reprendre l'initiative et à ne pas renoncer à faire entendre la voix de l'Europe. Nous sommes convaincus qu'il est encore temps d'éviter d'avoir et la guerre, et le déshonneur. Notre groupe votera donc cette proposition de résolution

La fin du califat, obtenue après un combat très dur où les FDS se sont illustrées par leur bravoure et leur détermination aux côtés de la coalition, n'a pas permis d'éradiquer totalement

personnes jetées sur les routes de l'exode, dans un pays qui compte déjà 6,6 millions de déplacés internes et 5 millions de réfugiés. En Syrie, plus de 50 % de la population est déjà réfugiée ou déplacée

dont dépendent pourtant à la fois notre sécurité, l'avenir du pays et la sécurité de ses voisins. Le condominium que cherchent à établir les trois pays du format d'Astana

Dans ce contexte mondial difficile et incertain, la France et l'Union européenne doivent être des puissances d'équilibre. Nous ne pouvons nous satisfaire d'être les vassaux des États-Unis ou de la Chine. Finalement, nous ne sommes Finalement, nous ne sommes pas des alignés. Il est important de pouvoir continuer à parler à tout le monde. La France, puissance d'équilibre, entend bien le faire. C'est ainsi que, dès le mois d'août, nous avons rehaussé notre dialogue avec la Russie, qui est désormais constant.

un peu frileux en matière de défense européenne et d'affirmation de notre autonomie stratégique. Il ne fait nul doute que le témoignage apporté par

Nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution. La conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explications de vote. Je mets aux voix la proposition de résolution.

Je voudrais entamer ce propos introductif en évoquant un exemple emblématique : en mars de cette année, une rave-party illégale a rassemblé près de 700 personnes à Lédenon, dans le Gard. Ce sont les habitants des villages des alentours, dérangés par les nuisances sonores à 2 heures du matin, qui ont alerté les gendarmes. La rave-party s'est tenue sur un terrain privé, sans autorisation préalable du propriétaire. Les gendarmes sont donc intervenus pour y mettre Les participants avaient emprunté des voies de défense des forêts contre l'incendie, exclusivement réservées aux sapeurs-pompiers, ce qui a engendré la détérioration de ces voies 160 conducteurs participant à cette fête y ont été verbalisés par les gendarmes. Sept infractions liées aux stupéfiants ont été relevées et trois pour des alcoolémies élevées. Surtout, la dégradation des lieux constatée le lendemain était éloquente : un terrain dévasté, des déchets partout et des résidus de drogues jonchant le sol. Devant la recrudescence de ces rave-parties, l'encadrement de leur pratique avait déjà été remanié en 2001, puis en 2002, par des textes venant modifier la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.

dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin, et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret. Les modifications prévoyaient notamment une déclaration officielle en préfecture pour les manifestations dont l'effectif prévisible dépasse 500 personnes, 500 personnes, devant être faite un mois avant la date prévue et assortie d'engagements pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publique. Des démarches sont à effectuer auprès des services de sécurité et de santé, des garanties devant être apportées sur le lieu choisi. Ces déclarations nécessaires et préalables ne sont pas effectuées la plupart du temps. Les maires des communes concernées m'alertent régulièrement sur l'existence d'une réelle problématique liée aux dégâts engendrés, selon la nature du site et l'importance de la manifestation.

menacent la biodiversité et entraînent des risques d'incendie, dans un contexte de sécheresse extrême. Rappelons que mon département, le Gard, figure parmi les départements les plus concernés à la fois par ces free-parties et par le risque de sécheresse. À l'heure où je vous parle, des mesures de restriction renforcées sont toujours en vigueur pour les usages de l'eau, malgré les premières précipitations importantes de l'automne. Même si les rave-parties ont généralement plutôt lieu au printemps et sont soumises aux interdictions au même titre que toutes les autres manifestations en période estivale,

Au-delà de ces nuisances environnementales, n'oublions pas la problématique des nuisances sonores pour les riverains. La question du bien-vivre ensemble, à laquelle je suis particulièrement attachée, doit également être évoquée, car, on le sait, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. le rappelle, l'objectif de cette proposition de loi n'est pas d'interdire une quelconque free-party ou de désigner des coupables, mais, au contraire, de susciter un débat apaisé et de mettre toutes les parties prenantes autour d'une table : les préfets, les maires, les organisateurs de rave-parties, les gendarmes, les associations de protection de l'environnement, les syndicats et les riverains concernés. Je souhaite que nous trouvions des solutions concertées pour mieux encadrer ces manifestations quand elles sont illégales et donner enfin les moyens aux communes, dont les maires apparaissent de plus en plus démunis face aux conséquences, d'exercer un pouvoir légitime sur le territoire dont ils ont la responsabilité et de préserver un environnement et une biodiversité de plus en plus menacés, comme l'actualité et les projets de loi que nous étudions nous le montrent chaque jour. Même si l'objectif premier de cette proposition de loi n'est pas de sanctionner de façon dogmatique et automatique, il apparaît que certains organisateurs, devant la légèreté des sanctions encourues, font fi des obligations J'ai donc souhaité introduire le débat en proposant un durcissement des sanctions frappant les organisateurs, dans la foulée des préconisations de la proposition de loi n° 864 déposée le 11 avril 2018 à l'Assemblée nationale par M. Thibault Bazin, député de Meurthe-et-Moselle. Comment renforcer ces pénalités ou sanctions pour dissuader l'organisation illégale et non déclarée de ces événements et comment ajuster la peine à la hauteur de l'infraction ? La question du mode de sanction, terme sans doute non approprié et à préciser lors des futurs débats, reste ouverte. Je me félicite des échanges constructifs que nous avons déjà eus avec le rapporteur à ce sujet à l'issue des différentes auditions. Les peines actuelles n'étant pas assez dissuasives, les rave-parties illégales continuent à perturber certaines régions avec leurs lots de conséquences néfastes : pour la santé des participants,

Mes chers collègues, il est nécessaire d'amorcer sur ce sujet un dialogue dépassionné et d'engager des mesures strictes pour encadrer l'organisation de ces événements quand ils sont illégaux. Il est également nécessaire de prévenir au mieux les nuisances et les conséquences sur l'environnement que les maires et leurs administrés doivent supporter.

mes chers collègues, la proposition de loi déposée par Mme Pascale Bories et plusieurs membres du groupe Les Républicains tend à résoudre un problème récurrent auquel les élus nationaux et les maires demandent, de longue date, une solution. Il s'agit, la réponse de l'État étant insuffisante, de mieux encadrer l'organisation de rassemblements festifs, généralement connus sous le nom de rave-parties, hors des lieux spécialement aménagés à cet effet, voire sans autorisation. Ces rassemblements appellent de la part des pouvoirs publics une attention particulière, du fait des troubles qu'ils peuvent susciter pour le voisinage, l'environnement et des dangers qu'ils comportent pour les participants. En l'état, le régime d'encadrement mis en place en 2002 ne fonctionne pas. Ce régime spécifique a transféré aux préfets les pouvoirs de police pour ce que les organisateurs appellent non plus des rave-parties mais des free-parties ou fêtes libres, qui sont qualifiées de « rassemblements exclusivement festifs à caractère musical » par l'article L. 211-5 de code de la sécurité intérieure. Ce régime, juridiquement très particulier, se présente comme un régime de déclaration, mais s'apparente en fait à un régime d'autorisation. Le préfet peut refuser de délivrer un récépissé et même interdire le rassemblement sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure. À l'inverse, le préfet doit engager une concertation avec les organisateurs si leur projet n'offre pas de garanties suffisantes. Cela peut le conduire à trouver un lieu pour l'organisation du rassemblement et à devenir en pratique coorganisateur de l'événement. Du fait de ce régime ambigu, il n'est pas étonnant que l'attitude de l'État ait oscillé entre des périodes d'appui aux organisateurs et des périodes de répression, pour se stabiliser aujourd'hui sur la base d'une tolérance de l'illégalité. En effet, de nombreux événements soumis à déclaration se tiennent alors même qu'ils n'ont pas été déclarés aux préfets ou qu'ils n'ont pas reçu de récépissé.

Au regard de cette situation, le nombre des condamnations est relativement faible, pour ne pas dire très faible ... Certains l'expliquent par le fait que la majeure partie des fêtes libres se passent bien, sans mise en danger des personnes et de l'environnement. Incontestablement, il y a, chez certains organisateurs et participants, un sens des responsabilités tout à fait louable. Toutefois, ces rassemblements restent de fait- parfois involontairement, souvent volontairement -hors la loi ; cette situation n'est pas tenable pour la sécurité des personnes et pour les maires qui en ont la charge au niveau des communes. paradoxalement, cet arsenal législatif et réglementaire comporte un angle mort. Pour concentrer les ressources des préfectures sur les rassemblements les plus importants, le régime d'encadrement actuel ne se déclenche qu'au-delà d'un seuil fixé par décret, qui est actuellement de 500 participants prévus. En deçà de ce seuil, c'est le maire seul qui doit gérer l'événement, mais comme aucune disposition spécifique n'est prévue, les fêtes libres de moins de 500 participants ne relèvent d'aucune police particulière et sont donc assimilées à de simples réunions.

en doublant la durée de saisie administrative du matériel et en transformant l'infraction de non-déclaration ou d'organisation malgré l'interdiction -actuellement une contravention de cinquième classe -en un délit. La commission des lois partage l'objectif des auteurs de la proposition de loi. Elle a cependant jugé qu'il n'était pas sûr, étant donné la réticence des services préfectoraux à mettre en oeuvre le dispositif actuel,

déclaration au maire. Cela lui permettra d'être informé et d'agir à temps, par la concertation ou, si nécessaire, par l'interdiction. En cas de non-déclaration ou d'interdiction, il sera possible de saisir le matériel ; ce n'est pas possible à l'heure actuelle pour les rassemblements de moins de 500 participants. Il s'agit là d'un régime de déclaration simple qui n'impose pas de nouvelles obligations aux maires. Nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de la discussion des amendements. S'agissant du renforcement des sanctions, la commission a considéré que la transformation de la contravention actuelle en un délit est une réponse adéquate et proportionnée au trouble que causent les rassemblements illégaux. La qualification en délit permettra désormais à la police judiciaire- gendarmerie ou police nationale -de conduire des enquêtes en flagrance, des interrogatoires, des perquisitions et des gardes à vue, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle. L'intention des auteurs de la proposition de loi est claire. Il s'agit non pas d'interdire les fêtes libres de musique techno parce qu'elles auraient une mauvaise image ou que ce genre de musique serait déplaisant, mais d'inciter les organisateurs à respecter le cadre légal, pour la sécurité des participants et le respect de l'ordre public, des populations et de l'environnement. Dès lors, plutôt qu'une peine de prison, qui ne serait de toute façon guère appliquée, la commission a prévu, comme c'est le cas pour les dégradations visées à l'article L. 322-1 du code pénal, que la peine encourue pour le nouveau délit soit une amende de 3 750 euros et des travaux d'intérêt général dont la durée maximale serait de 400 heures, soit 53 jours de travail effectif, contre 120 heures au plus à l'heure actuelle. La rédaction de l'article relatif à la requalification en délit a également été précisée afin d'être pleinement conforme au principe de légalité des délits et des peines et de permettre la confiscation des biens saisis. Par ailleurs, la commission n'a pas retenu le doublement de la période de saisie administrative envisagé dans la version initiale de la proposition de La commission a enfin souhaité que l'on puisse fournir un appui au maire dans son dialogue avec les organisateurs et, si possible, sortir de la situation actuelle de blocage au niveau de l'État, qui aboutit à la tolérance de l'illégalité. Afin de relancer le dialogue entre les pouvoirs publics et les organisateurs, qui disent vouloir entrer dans la légalité et démontrer leur sérieux, la commission souhaite qu'une charte de l'organisation de ces rassemblements soit définie par les pouvoirs publics après négociation avec les organisateurs. Ceux qui y adhéreront feront la preuve de leur engagement à respecter la loi, ce qui facilitera leur dialogue avec les maires et les préfets. Le régime des fêtes libres a vocation à se fondre dans le régime général des spectacles, festivals et événements culturels, mais les organisateurs de ces rassemblements restent aux marges du droit. Il s'agit de permettre à ceux qui souhaitent rentrer dans la légalité de le faire, de sanctionner les autres et, surtout, de redonner aux maires les moyens d'agir pour la sécurité des personnes,

les sénateurs, c'est un point auquel le Gouvernement est attaché. Nous croyons que les maires sont l'un des maillons les plus essentiels de la République ; le projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, que

d'un amendement allant dans le bon sens. La mesure principale du texte consiste à créer un régime de déclaration auprès du maire pour les rassemblements festifs à caractère musical devant compter moins de 500 participants. Cette mesure pose un certain nombre de difficultés. D'abord, elle crée un régime de police spéciale concurrent à celui du préfet pour les rave-parties, sans pour autant l'assortir de pouvoirs de police dédiés, comme ceux dont disposent les préfets en la matière.

Ainsi- je le dis comme membre du Gouvernement, mais aussi comme ancien préfet, et donc praticien -, cette mesure risquerait d'avoir des effets pervers dommageables. Pour éviter que le préfet fasse usage de ses pouvoirs de police spéciale, les organisateurs de rave-parties pourraient être tentés de volontairement sous-évaluer l'affluence

Ensuite, je pense qu'il est important de rappeler que les rave-parties se tiennent souvent sur le territoire de petites communes, qui pourraient être dépassées par les demandes : elles n'auraient pas suffisamment de marges de manoeuvre et de ressources pour préparer les rassemblements et en assurer efficacement la protection. protection. Dépassées, ces petites communes pourraient également être amenées à solliciter l'appui du préfet ou sa substitution du fait de leur carence, pour des événements dont l'ampleur n'aurait potentiellement pas justifié un investissement lourd de la préfecture.

Deux raisons me poussent à émettre certaines réserves sur ce point. D'abord, l'existence d'une telle charte relève non pas du pouvoir législatif, mais du pouvoir réglementaire. Ensuite, cette charte existe déjà : elle est prévue par l'article R. 211-8 du code de la sécurité intérieure et son contenu a été fixé dans un arrêté du 3 mai 2002. Enfin, la dernière partie de ce texte crée un nouveau délit qui se substitue à la contravention de cinquième classe actuellement prévue en cas de non-respect des obligations de déclaration.

général. Si nous pourrions être favorables à la création d'un délit sanctionnant le non-respect d'une obligation de déclaration d'un grand rassemblement, afin de réprimer l'impossibilité faite aux autorités d'anticiper et de protéger, nous ne pouvons l'être quand il s'agit de sanctionner le non-respect d'une obligation portant sur des rassemblements de faible envergure, ce à quoi le texte de la proposition de loi aboutit. De même, pour assurer une répression efficace,

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l'aurez compris, si le Gouvernement partage sans ambiguïté les objectifs sous-tendant cette proposition de loi, ainsi que la volonté de Pascale Bories et de Henry Leroy de donner plus de pouvoirs aux maires, le texte examiné aujourd'hui nous oblige aux plus grandes réserves.

Accompagnant la révolution numérique et détrônant la culture du rock, cette musique a conquis l'Europe par le phénomène des rave-parties. Souvent clandestines, ces soirées investissent des endroits isolés, comme des hangars, des carrières ou des champs, au grand dam des élus et des habitants de nos territoires ruraux qui voient leurs villages tranquilles envahis par des hordes de jeunes fêtards. Ces manifestations, qui se déroulent indifféremment dans des propriétés publiques ou privées, ont été le théâtre de drames ; certains incidents graves ont émaillé ces rassemblements clandestins. Qu'il s'agisse d'alcool, personne n'est dupe quant à l'usage de stupéfiants dans ces soirées, qui occasionne parfois des décès ou des incidents sanitaires graves. Lorsque, dans le meilleur des cas, aucune victime n'est à déplorer, c'est l'environnement même de la manifestation qui subit des dommages.

certains maires prennent des arrêtés d'interdiction, ils sont malheureusement incapables d'en assurer l'effectivité. Spectateurs désabusés, les maires attendent l'intervention des services de l'État. Un dispositif spécifique a bien été mis en place en 2002 pour l'encadrement des rassemblements exclusivement festifs à caractère musical. Il a rapidement montré ses limites : en pratique, il ne permet pas de faire entrer les organisateurs dans la légalité. Par ailleurs, le maire est seul pour gérer les rassemblements de moins de 500 participants. Enfin, ce dispositif est paradoxal, monsieur le secrétaire d'État. Actuellement, il est plus facile d'organiser une fête libre qu'une activité artistique amateur Organisées sur des terrains privés, ces fêtes libres, qui relèvent du régime des réunions, requièrent la seule autorisation du propriétaire. Au contraire, le moindre spectacle amateur doit faire l'objet d'une déclaration au maire de Mme Bories prévoit d'abaisser le seuil qui déclenche l'obligation de déclaration au préfet. Il double la durée de saisie administrative du matériel. L'infraction de non-déclaration ou d'organisation malgré l'interdiction, simple contravention de cinquième classe, devient un délit ; c'est important. Au cours de ses Au cours de ses travaux, la commission a toutefois préféré ne pas modifier le seuil qui détermine la compétence du préfet. Elle a renforcé les moyens dont disposent les maires pour faire face à ce type de rassemblements. Ceux de moins de 500 participants devront dorénavant obligatoirement être déclarés aux maires. Afin de permettre aux organisateurs de faire la preuve de leur capacité à organiser un rassemblement respectant l'ordre la tranquillité publique et l'environnement, la commission a également prévu l'élaboration d'une charte, dont le contenu sera défini par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse après concertation avec les représentants des organisateurs. Enfin, personnellement, je regrette un peu que la commission des lois- Dieu sait

Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, approuvant l'excellente démarche de notre collègue Mme Bories,

et des différentes mesures proposées, une question m'est venue à l'esprit : pourquoi certaines de celles-ci n'ont-elles pas été intégrées dans ce texte d'origine gouvernementale, qui a sans doute plus de chances de prospérer que la présente proposition de loi ? Je regrette d'ailleurs qu'un certain nombre de nos propositions de loi ne soient pas reprises

Le débat en commission, mercredi dernier, a été nourri ; il a permis de repenser le régime d'encadrement de ces rave-parties, appelées aussi free-parties, ou fêtes libres. Il s'agit d'un problème auquel les élus et, plus spécifiquement, les maires sont confrontés de manière récurrente, sans que de nouvelles solutions soient proposées. Ces rassemblements festifs se déroulent le plus souvent hors des lieux spécialement aménagés à cet effet, ce qui entraîne des dégradations. Comme cela a été rappelé, le dispositif actuel repose sur la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, qui a connu au fil des ans quelques modifications :

Cependant, on ne peut que constater l'extrême ambiguïté de ce régime juridique. Présenté comme une simple obligation de déclaration par les organisateurs, il s'apparente en réalité à un régime d'autorisation, le préfet pouvant refuser de délivrer le récépissé, voire interdire le rassemblement. À l'inverse, le préfet doit engager une discussion avec les organisateurs dans le cas où le projet n'offre pas les garanties suffisantes et « alors tenter d'adapter les mesures prévues et, le cas échéant, rechercher un local ou un terrain plus approprié ». Autrement dit, le préfet s'apparente à un co-organisateur de l'événement.

Notre rapporteur a rappelé que, en 2018, pour 800 rassemblements qui auraient dû être déclarés, seulement deux récépissés auraient été délivrés par les préfets. La plupart de ces fêtes se sont donc déroulées sans autorisation ni, évidemment, concertation préalable. Les sanctions encourues sont peu dissuasives- une contravention de cinquième classe et, éventuellement, la confiscation du matériel utilisé -et n'incitent pas les organisateurs à faire une déclaration en préfecture. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les maires se trouvent démunis pour gérer les rassemblements de moins de 500 participants ; les organisateurs doivent simplement demander l'autorisation du propriétaire du terrain où ils souhaitent tenir leur fête. Cet après-midi, mes chers collègues, il s'agit de renforcer le pouvoir des maires en matière de rave-parties et de renforcer le cadre légal de ces manifestations. C'est l'objet de la principale modification qu'a apportée notre commission des lois à l'article 1 de cette proposition de loi,

Henri Leroy, et visant à renforcer l'encadrement des rave-parties et les sanctions à l'encontre de leurs organisateurs. L'article 1 remanié étend l'obligation de déclaration des organisateurs auprès des maires, au moins un mois avant la date prévue, aux rassemblements de moins de 500 personnes. La déclaration devra détailler les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. L'article 1 , introduit sur l'initiative du rapporteur, prévoit une charte de l'organisation de ces rassemblements. L'article 2 étend aux maires la possibilité de saisie des matériels et substitue au prononcé d'une peine de prison la possibilité de décider d'un travail d'intérêt général. Le rapport de M. Leroy établit une bonne synthèse des paradoxes que nous rencontrons souvent dans notre

dispositif qui permet en réalité d'empêcher la tenue d'un événement, mais je ne veux pas croire que ce soit ici la volonté de la majorité sénatoriale ! M. Leroy nous donne des chiffres intéressants sur le nombre de rave-parties organisées dans notre pays.

le nombre de condamnations paraît faible. D'après les éléments communiqués à votre rapporteur, il y aurait 70 condamnations par an à la contravention prévue par l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure, pour un montant de 418 euros en moyenne. Ce montant apparaît relativement élevé par rapport au montant maximal encouru lorsqu'on le compare à celui des amendes prononcées pour d'autres contraventions, mais il demeure faible dans l'absolu. La peine complémentaire de confiscation du matériel n'est pour sa part prononcée qu'en moyenne deux fois par an.

en termes de nuisances sonores, voire de dégâts causés à l'environnement ou aux terrains utilisés. Je m'interroge néanmoins sur l'opportunité de cette proposition de loi : le péril est-il si immense que nous devions de nouveau durcir la loi ?

Il faut se méfier des nouveaux pouvoirs donnés aux maires quand les moyens de les mettre en oeuvre ne suivent pas. De nombreux maires risquent de se retrouver tiraillés entre, d'un côté, des riverains opposés à des rave-parties perçues uniquement comme des nuisances, et, de l'autre, des organisateurs de bonne foi- il y en a aussi ! -fatigués de devoir toujours se justifier davantage. M. le président de la commission a relevé nos divergences. Oui ! J'ai peur que le changement de philosophie sous-tendant la réglementation sur les rave-parties ne pousse davantage d'organisateurs vers la clandestinité, mais je peux comprendre que les craintes d'un évitement de la loi ne suffisent pas à justifier un refus d'évolution de la législation. Je soulignerai cependant que le public des rave-parties, qui ne se caractérise pas toujours par son adhésion aux institutions, ... C'est une litote ! ... se révèle souvent particulièrement imaginatif en matière de contournement de la loi. Par ailleurs, je ne voudrais pas que l'on considère les rave-parties comme néfastes par nature. Mon département connaît peu de rassemblements d'envergure. Aux dires des organisateurs que j'ai contactés, notre géographie décourage beaucoup de promoteurs d'événements : il est selon eux difficile de trouver des terrains suffisamment éloignés des habitations pour organiser des événements en toute tranquillité.

est aujourd'hui un ambassadeur de la musique française dans le monde et a été fait chevalier de la Légion d'honneur. Nous devons trouver un équilibre pour ne pas réprimer les Laurent Garnier de demain, tout en nous assurant que les rave-parties ne gênent pas plus de monde qu'elles n'en satisfont.

au moment où nous examinons la proposition de loi de nos collègues du groupe Les Républicains visant à mieux encadrer les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, je souhaite rappeler que l'attrait ancestral socioculturel et l'attrait plus contemporain économico-touristique de la fête dans notre société ne sont plus à démontrer. Il n'est pas question aujourd'hui d'interdire des manifestations festives, par définition transgressives ; il s'agit bien plutôt de réfléchir aux moyens de permettre leur déroulement en toute sécurité. C'est le coeur de la proposition de loi que nous discutons aujourd'hui. Dans nos territoires, les festivals, les carnavals et plus particulièrement, dans ma région, les férias rythment l'année. Ces événements festifs, qui peuvent être perçus comme des rassemblements transgressifs à visée cathartique, sont en réalité des faits sociaux, normés et formalisés par la coutume. Ce que l'on a appelé, à partir des années quatre-vingt-dix, les rave-parties, puis les free-parties, sont par définition des rassemblements exclusivement festifs à caractère musical qui rejettent les normes coutumières de la fête traditionnelle. Ils constituent une part de la scène musicale « underground », une offre culturelle en marge des événements musicaux organisés par des institutions culturelles reconnues et des établissements de fêtes nocturnes. Si elles échappent à toute logique commerciale et se définissent par leur accessibilité et leur spontanéité, les rave-parties se caractérisent aussi par leur organisation anarchique, leur localisation inattendue et, parfois, des commerces illicites. Pour toute personne attachée comme moi au respect de l'ordre public et à la protection du droit de propriété, la première préoccupation, s'agissant des free-parties, est de s'assurer que leur tenue n'y porte pas atteinte, tout en exigeant qu'elles ne mettent en danger ni les participants ni les riverains.

Ces considérations ont d'ailleurs été à l'origine de l'adoption du dispositif Vaillant, fixant en 2001 un premier régime d'encadrement des rave-parties. Les services de l'État ont la responsabilité de l'encadrement des rassemblements de plus de 500 personnes, seuil défini par décret, décret, les préfets agissant en concertation avec les maires et les organisateurs. D'après le délégué ministériel à la jeunesse, sur 800 rave-parties de plus de 500 personnes organisées en 2018, seulement deux ont été interdites. En règle générale, ces événements ne sont pas interdits lorsqu'ils sont régulièrement déclarés en préfecture. Le dispositif Vaillant pourrait donc fonctionner, s'il était appliqué systématiquement. Pour les rassemblements regroupant plus de 500 personnes, la préfecture tend à mobiliser les forces de l'ordre pour assurer l'encadrement, avec une certaine tolérance. Toutefois, comme le pointent les auteurs de la proposition de loi,

Le rapporteur nous a informés qu'il s'agissait d'un phénomène particulièrement présent dans le Sud-Ouest, où se déroulerait la majorité des 3 200 free-parties de moins de 500 personnes dénombrées sur le territoire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas seulement de rassemblements en zones rurales : les zones semi-urbaines et urbaines sont également touchées. J'ai eu à tenter de gérer des free-parties dans les friches industrielles de la métropole bordelaise Pour les maires, chargés de prévenir tout trouble de voisinage sans toutefois endosser la responsabilité des risques liés à ces rassemblements, le régime actuel n'est pas satisfaisant, car il les place en première ligne pour la négociation avec les organisateurs, sans leur conférer de moyens de police suffisants pour empêcher, Si certains maires ne souhaitent pas avoir à gérer ces free-parties, nous devons entendre la position des maires qui, pour protéger les participants à ces fêtes, sont favorables à l'organisation de tels rassemblements festifs sur le territoire de leur commune. Lorsque ces rassemblements ne dérangent personne et ne portent pas atteinte à la propriété d'autrui, pourquoi les interdire ? Henri Cabanel a beaucoup travaillé sur cette problématique et sa contribution à la réflexion a été précieuse. Free-party signifie fête à la fois libre et gratuite

à l'égard de ces événements. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les amendements que je défendrai tout à l'heure. Ils visent respectivement à associer les maires à la rédaction de la charte proposée par le rapporteur, à ne pas mettre à leur charge la confiscation du matériel et à instaurer une coresponsabilité entre les maires et les préfets pour garantir la sécurité autour des rassemblements de moins de 500 personnes. Il s'agit de permettre aux maires d'informer et de mobiliser les préfets lorsqu'ils constatent l'impossibilité pour

Nous en sommes conscients, sans pour autant vouloir nous enfermer dans une rhétorique hostile à ces festivités ou à ces genres de musique qui recherchent la transcendance et expriment une forme de refus du mercantilisme.

sous-tendant ce texte, tels qu'ils ont été repris à son compte par la commission des lois, sur proposition du rapporteur. Oui, nous voulons permettre à ceux qui souhaitent entrer dans la légalité de le faire. Oui, nous voulons aussi sanctionner le plus intelligemment possible lorsque les circonstances de l'espèce le justifient.

coexistence de deux régimes de police spéciale. Comment mettre en application ce pouvoir de police lorsque l'on est tributaire des possibilités d'intervention des forces locales de sécurité ?

on aboutit, par suite logique, à deux régimes de police spéciale identiques, relevant pour l'un du maire, pour l'autre du préfet, avec pour seul critère discriminant le nombre prévisible de participants,

par des personnes qui bafouent ouvertement la loi avec la bénédiction des pouvoirs publics, on doit être beaucoup plus restrictif et dissuasif.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la lecture de cette proposition de loi a rappelé à mon souvenir un certain nombre de textes du même acabit

de la commission des lois, qui a substitué à la peine de prison une peine de travail d'intérêt général. Cela est heureux, car le texte de la proposition de loi initiale était symptomatique d'une dérive maintenant beaucoup trop fréquente, qui conduit à légiférer au moindre fait divers, en proposant des durcissements de notre code pénal, en considérant que dissuader passe nécessairement par la relecture de notre code pénal, en jugeant que la contravention, même de cinquième classe, n'est rien au regard des délits et des peines d'emprisonnement,

Comme l'indique le président de l'association Technopol, Tommy Vaudecrane, durcir les sanctions ne sert à rien : « il vaut mieux s'entretenir avec les responsables ». D'ailleurs, selon lui, lors de ces rassemblements, « il n'y a pas plus d'accidents que dans les férias, les sorties de boîte de nuit, les soirées étudiantes ou tout autre événement légal. [ ...] On balance le tout-sécuritaire pour faire peur aux gens, alors que beaucoup d'événements sont autogérés et gèrent bien les incidents.

Il s'agit là, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, d'une mesure plutôt acceptable, bien qu'elle n'engage pas à grand-chose. Pour le reste, selon nous, l'encadrement législatif et réglementaire déjà existant rend tout nouveau dispositif législatif inutile. En effet, les « rassemblements festifs à caractère musical » sont déjà largement encadrés. La loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité en a fait mention pour la première fois,

d'organiser une concertation avec les responsables pour adapter lesdites mesures d'encadrement ou rechercher un terrain ou un local plus approprié. Pour nous, transférer ces pouvoirs au maire n'est pas la solution, comme nous avons eu l'occasion de le souligner lors de la discussion du projet de loi Engagement et proximité, que nous venons d'adopter. concerne les impacts de ces rassemblements festifs sur la biodiversité, nous ne pouvons bien sûr rester insensibles à cette question préoccupante, mais force est de constater que le texte ne l'évoque qu'à la marge.

Quelle que soit l'appellation de ce qui pourrait apparaître comme un avatar du « droit à la fête »- rave-party ou free-party -, la recrudescence de ce phénomène conduit à traiter des questions qui touchent à l'atteinte à des droits aussi essentiels que le droit de propriété, avec en contrepoint l'occupation sauvage de terrains publics ou privés, le droit à la préservation de l'environnement, avec en contrepoint des atteintes à la biodiversité lors des occupations sauvages, ou le droit à la santé, avec en contrepoint des trafics de substances incontrôlées

de déclaration ou le non-respect de l'interdiction préfectorale ne sont passibles que d'une contravention de cinquième classe, éventuellement assortie d'une saisie du matériel utilisé pour une durée maximale de six mois, on mesure facilement les limites du dispositif de contrôle et l'inanité du système actuel. On comprend aussi que nombre d'organisateurs de rave-parties ricanent devant la légèreté des sanctions encourues. Ces dernières n'étant pas assez dissuasives, les rave-parties illégales fleurissent à travers nos régions, avec leur lot de débordements. Malheureusement, il est courant que des incidents graves émaillent ces rassemblements clandestins.

En 2016, un jeune de 20 ans a trouvé la mort en marge d'une rave-party organisée à Saint-Antonin-Noble-Val. Nuisances sonores assourdissantes, terrains dévastés, comas éthyliques et overdoses, atteintes sexuelles, dévastation des lieux : tel est le lot de bien des rave-parties organisées de façon illégale.

Force est donc de constater que le régime juridique actuel se révèle peu efficace pour faire entrer l'organisation de ces rave-parties dans la légalité, pour garantir la sécurité de leurs participants, la protection de l'environnement et la tranquillité des riverains.

afin de permettre à ces derniers de prendre les mesures nécessaires lorsqu'une rave-party doit se tenir sur le territoire de leur commune. De même, la possibilité de saisie du matériel en cas de méconnaissance de leurs obligations par les organisateurs peut permettre une véritable efficacité opérationnelle, qui manque aujourd'hui. Enfin, nous avons conclu à la nécessité de renforcer les sanctions en prévoyant la création d'un délit assorti d'une peine de travail d'intérêt général. L'objectif est non pas d'interdire les « teufs

chaque année, plus de 3 200 rave-parties sont organisées en France, majoritairement dans des zones rurales, presque toujours sur des terrains privés, sans qu'aucune autorisation ait été demandée par les organisateurs. En 2015, lorsque j'étais directeur des études de l'Institut d'études judiciaires, j'avais demandé à la gendarmerie de venir faire de la prévention auprès de mes étudiants.

voitures avec groupe électrogène, caméras, patrouilles cynophiles ... -pour garantir la sécurité des personnes et des biens aux alentours du site, limiter les nuisances pour les riverains

La gendarmerie devait aussi garantir la fluidité de la circulation en périphérie de la zone, grâce à la présence d'unités de force mobile sur le terrain. La préfecture avait mis en place des supports logistiques pour l'eau, l'électricité, les sanitaires. Une zone de soins avait été installée, avec des lits d'appoint et des tentes. Une clôture avait même été dressée autour de l'emprise de la zone du Teknival pour délimiter la manifestation. À l'issue de cette présentation, tous mes étudiants

stricte et généralisée, compte tenu des risques qui existent à plus ou moins grande échelle. Notre objectif n'est pas bien sûr d'interdire ces rassemblements. Nous devons simplement prendre les mesures nécessaires pour faire respecter les lois et l'ordre public.

Dans un état de droit, où la liberté reste la règle, les organisateurs doivent simplement prendre leurs responsabilités en trouvant un lieu adéquat, en concertation avec les pouvoirs publics, afin d'occasionner le moins de gêne possible en facilitant la mission d'accompagnement, de sécurisation et de maintien de l'ordre public des gendarmes ; en remettant en état le site sur lequel s'est déroulé le rassemblement. Seul un dialogue constructif est en mesure d'apporter les garanties nécessaires. Aujourd'hui, la loi prévoit que c'est au maire qu'il appartient de gérer ces événements lorsque les rassemblements n'excèdent pas 500 participants. Or, comme je l'ai dit plus tôt, ces rassemblements ayant généralement lieu dans des zones rurales peu habitées, les maires sont trop souvent démunis. Ils disposent de moyens trop faibles pour appréhender ces réunions.

La commission des lois a exploré la possibilité de mettre en place une charte de l'organisation des rassemblements, qui serait définie, après négociation avec les organisateurs, par les pouvoirs publics. Je salue cette initiative, qui me semble aller dans le bon sens. Nous ne pouvons pas empêcher toutes les rave-parties de se tenir. Ce que nous pouvons faire, en revanche, c'est inciter les organisateurs à rester dans la légalité. C'est l'objectif de cette proposition de loi. À cet égard, il convient d'ailleurs de préciser que nombre de ces rave-parties se déroulent dans une atmosphère bon enfant.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, « les raves-parties à répétition exaspèrent », « on en a marre », « on n'en peut plus » : voilà ce que nous entendons trop souvent.

problèmes : une circulaire a alors mis l'accent sur la vente et la consommation de stupéfiants. Une autre, en 1998, a distingué, d'une part, les organisateurs effectuant une demande auprès des services administratifs, et, d'autre part,

seules sept raves ont été déclarées dans mon département de l'Eure, puis neuf en 2003. Or nous connaissons tous la réalité dans nos territoires : nous savons tous qu'il y en a bien plus, dans l'Eure comme ailleurs. Il est évident qu'une grande partie de ces événements

est aujourd'hui l'objet de ce texte, qui vient à point pour étendre le champ des déclarations préalables et donner le contrôle de celles-ci aux maires pour les événements rassemblant moins de 500 participants. D'abord, il faut ouvrir les possibilités d'agrément pour les organisateurs, afin qu'ils ne soient plus tentés de passer outre la déclaration préalable et d'organiser des raves illégales. Ce texte y parvient avec brio.

En outre, les rave-parties rassemblent des participants venus parfois de loin et prévenus longtemps en avance sur les réseaux sociaux. La communication s'organise en effet au mépris de la loi, par le maintien d'une imprécision sur le lieu de rendez-vous, souvent en le modifiant à la dernière minute. Il convient donc d'encadrer ce canal, en ne permettant pas la diffusion d'informations sur la tenue d'une rave avant l'agrément

et 102 décibels sur quinze minutes. Le niveau sonore est une nuisance, pour ne pas dire « la » nuisance principale, tant pour les participants que pour le voisinage. Il est essentiel qu'il soit connu. Il faut donc inciter les organisateurs à installer des écrans affichant en direct le volume diffusé, de la même manière que dans les festivals. Notre rôle sera désormais de rester attentifs à la mise en oeuvre de cette proposition de loi, en particulier concernant le périmètre des éléments mentionnés par les organisateurs et la réponse des maires lorsqu'une rave se tient sur les territoires limitrophes de plusieurs communes. Je voterai cette proposition de loi.

C'est vrai qu'il faut encadrer ce genre de festivités, qu'il faut trouver des solutions, mais on ne peut pas empêcher les débordements. C'est la partie économiquement libérale du Sénat qui a élaboré ce texte. qui a élaboré ce texte. Le festival de Woodstock n'a pas empêché les États-Unis de demeurer le champion du libéralisme économique ! C'était pourtant le temple du sexe, de la drogue, de Jimi Hendrix, etc. etc. M. Bas n'était pas encore né à cette époque ! Je persiste à dire que ces fêtes sont des soupapes de sécurité pour la société. M. Bas me dira que c'est de la philosophie, mais il faut bien un peu de philosophie pour gérer les sociétés, pas seulement

L'article 1 prévoit l'information préalable des maires avant tout rassemblement, via un nouveau régime de déclaration, pour tous les cas où le préfet n'est pas compétent, notamment lorsque moins de 500 personnes sont attendues et en l'absence de publicité. Quelle que soit la taille du rassemblement, les organisateurs devront désormais présenter les documents permettant d'organiser précisément le rassemblement. De ce point de vue, le texte me semble être une avancée. J'ajouterai juste à l'adresse de notre collègue Benbassa, avec qui nous avons souvent l'occasion de discuter de ces sujets, que j'ai apprécié sa culture politique, ses références à Woodstock, naturellement,

Toute limite à ce droit serait forcément de nature autoritaire. Je pense qu'il faut resituer un peu les choses. Ces personnes ne supportent pas la moindre contrainte formaliste permettant d'organiser au mieux ces événements plutôt que de les subir.

parole est à M. Jérôme Durain. Les rave-parties sont régies par le code de la sécurité intérieure, dans sa partie législative, ainsi que dans sa partie réglementaire. Ces manifestations sont donc précisément encadrées. D'une part, il existe les dispositions générales qui relèvent de la loi. D'autre part, les formalités pratiques auxquelles doivent se soumettre les organisateurs de rave-parties sont renvoyées au domaine réglementaire. En prévoyant une nouvelle déclaration auprès du maire pour tous les cas où le préfet n'est pas compétent, l'article 1 crée un nouveau régime déclaratif. La volonté de donner aux maires la capacité d'anticiper pareille manifestation est légitime. L'esprit de dialogue et d'accompagnement qui a présidé à l'élaboration du cadre législatif en vigueur pour les rave-parties de taille importante serait ainsi appliqué aux rave-parties de moyenne importance. Afin d'assurer la cohérence de l'ensemble des dispositions relatives aux rave-parties, l'amendement que nous présentons vise simplement aligner le régime destiné aux « petites » raves sur le régime en vigueur. En effet, la précision relative au délai d'un mois est de nature réglementaire. Il serait approprié de laisser le décret définir cette durée, au même titre que pour les grands rassemblements. Je rappelle que lorsque nous avons porté en 2006 de 250 à 500 le nombre de participants à partir duquel une déclaration est rendue obligatoire afin de mieux cibler les gros événements qui préoccupaient alors les pouvoirs publics, cette précision étant de nature réglementaire, un simple décret du ministre de l'intérieur Nicolas Sarkozy a suffi. Il n'a nullement été besoin de légiférer. Je signale au passage que nous aurions également pu demander la suppression de l'alinéa 4 de l'article 1, qui impose de mentionner dans la déclaration les nuisances de toutes natures qui peuvent résulter

pour les regroupements supérieurs à 500 personnes. Or, en Gironde par exemple, ce sont surtout de plus petits rassemblements qui sont organisés, sous forme de free-parties. Dans ces situations, nous l'avons tous évoqué ici,

dans des conditions susceptibles de satisfaire les participants, les riverains et les conditions de sécurité, ils ne peuvent là aussi parfois compter que sur eux-mêmes pour mobiliser les forces de l'ordre et la préfecture. Cet amendement tend donc à mettre en place un régime de responsabilité partagée entre les maires et l'État, les maires ayant la charge de la concertation et de l'information, les services de la préfecture celle de l'intervention, si nécessaire, afin de garantir la sécurité de ces manifestations. Quel est l'avis de la

Surtout, l'amendement fait référence à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités locales, qui prévoit que le préfet peut se substituer aux maires défaillants pour assurer la salubrité, la sûreté, la tranquillité publique. Il est difficile d'écrire dans la loi que le maire peut invoquer sa propre carence pour faire intervenir le préfet.

monsieur les rapporteurs,

Les forces de gendarmerie sont particulièrement mobilisées pour sécuriser les lieux. Il apparaît donc logique dans ce cas de mettre à la charge des organisateurs les frais liés aux services d'ordre effectués au-delà des obligations normales incombant à la puissance publique. Dans une vie antérieure, monsieur le secrétaire d'État, j'ai été élu dans le Larzac.

qui permet l'information du maire un mois avant la tenue d'un rassemblement, mais il ne lui confère pas de nouveau pouvoir de police, donc pas d'obligation supplémentaire.

Depuis 1981, le ministère de la culture a connu des évolutions importantes dans l'exercice de ses missions, et la notion de culture s'est considérablement élargie. Des formes d'expression jugées mineures ou réservées à certaines catégories sociales considérées comme plus ou moins marginales ont été reconnues comme légitimes. La musique techno est aujourd'hui bien identifiée comme une expression musicale à part entière qui mérite l'attention des pouvoirs publics. La production de la musique électronique se réinvente au gré de l'évolution des nouvelles technologies. En matière économique, elles représentent 17 % des musiques actuelles. On aurait donc pu imaginer une implication importante du ministère de la culture sur la question des raves-parties. Force est de constater une situation inverse. Depuis le début, nous avons bien assisté à un phénomène de captation de ce problème par le ministère de l'intérieur et la mise à l'écart du ministère de la culture. Ce désengagement quasi total du ministère de la culture est une anomalie. Un tel processus n'est pas sans effet sur la manière d'aborder le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. La remise en jeu du ministère de la culture n'est donc pas neutre. Dans certains cas, ce ministère a joué un rôle de médiation utile entre les groupes de musique électronique animant les raves et les autorités politiques. Nous pouvons citer en exemple ce qui se passe en Bretagne et dans la région limitrophe des Pays de la Loire. Bien avant la charte visée par l'article 1 de la proposition de loi, des livrets à l'usage des démarches de concertation ont été élaborés. Dans ces territoires, qui sont les plus vivants en matière de rave-parties et qui ont été des terrains d'affrontements violents entre les forces de l'ordre et les « teufeurs », l'engagement du ministère de la culture et d'une multitude d'acteurs culturels publics et associatifs démontre qu'une autre voie est possible pour traiter la question des rave-parties. Quel est l'avis de la

Je voudrais remercier M. le rapporteur, qui a compris tout l'intérêt qu'il y avait à associer le ministère de la culture : plus il y aura de parties prenantes autour de la table et plus on arrivera à trouver des solutions.

Comme l'a souligné notre collègue Henri Cabanel, un guide de la médiation avait jadis été rédigé en interministériel, sous le pilotage du ministère de la jeunesse de l'époque, en dialogue avec un panel d'organisateurs. Il serait efficace que cette charte s'inspire de ces travaux antérieurs, ces derniers ayant permis quelques avancées sur le terrain.

il n'est pas très cohérent d'avancer que l'on souhaite coopérer en amont avec les organisateurs et, dans le même temps, les mettre sous répression pénale en transformant la contravention en vigueur en délit. Les organisateurs savent très bien que le régime de la déclaration est un régime d'autorisation déguisée. La pratique a suffisamment démontré cette réalité. Pareille option, si elle venait à être retenue par le Sénat, risquerait de se retourner contre les élus locaux. Comme ils auront tendance à considérer que les conditions ne sont pas suffisamment réunies, ils pourront s'y opposer. Or notre rapporteur a rappelé à plusieurs reprises que le présent texte ne créait aucun pouvoir de police du maire. Ce texte n'instaure qu'un régime de déclaration simple sans possibilité de refuser

la manifestation éprouveront le sentiment qu'en jouant le jeu du régime déclaratoire ils risquent de se faire piéger davantage, ils ne pourront qu'être incités fortement à choisir la clandestinité. La question porte essentiellement sur les petites raves. Nous ne disposons pas de statistiques précises pour connaître l'ampleur du phénomène. Notre rapporteur a rappelé que les enquêtes connues sont anciennes et les chiffres peu fiables. Nous légiférerons donc à l'aveugle alors qu'il existe déjà

Au contraire, ainsi que l'exprime le Conseil d'État, qui dénonce régulièrement les effets de l'intempérance normative, ce serait source d'instabilité et de complexité, et, sur le terrain, cela pourrait bien de se retourner contre les maires. Face à leur sentiment d'isolement et l'incapacité d'agir, les maires demandent au contraire à être mieux entendus et mieux accompagnés dans leurs pouvoirs de police lorsque des rassemblements festifs à caractère musical sont organisés sur le territoire de leur commune. Quel est l'avis de la ? Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de pouvoir de police du maire ; j'ai dit qu'il n'y avait pas de pouvoir « spécial » de police du maire ! La situation actuelle, qui réprime l'interdiction des manifestations par une contravention de cinquième classe, a fait la démonstration de son incapacité à fonctionner. Le fait de le passer en délit donne des pouvoirs aux services de police et de gendarmerie pour faire respecter la règle. Aujourd'hui, tout est bloqué. Comme cela a été rappelé, 3 200 manifestations ne nécessitent pas de déclaration aux préfets,

Mme Nicole Duranton. La lutte contre l'organisation de rave-parties sauvages doit passer par des prévisions de sanctions à même de dissuader effectivement les organisateurs potentiels de ces événements. Cet amendement vise donc à augmenter l'amende prévue sans pour autant la rendre équivalente aux peines encourues pour des faits plus graves.

Les rave-parties réunissent des participants venant parfois de loin et prévenus longtemps en amont sur les réseaux sociaux. La communication sur celles-ci s'organise en effet au mépris de la loi par le maintien d'une imprécision sur le lieu de rendez-vous, souvent en le modifiant à la dernière minute. Il convient donc d'encadrer ce canal, en ne permettant pas la diffusion d'informations sur la tenue d'une rave avant l'agrément préfectoral ou municipal.

du principe de légalité des délits et des peines. En l'état, cela pourrait toucher non seulement les organisateurs, mais aussi la presse et des autorités publiques elles-mêmes. Cet amendement risque donc de ne pas atteindre sa cible. De manière plus pratique, c'est aux pouvoirs publics quand ils de rendre la décision publique. Il convient que les maires soient appuyés par les services de police et de gendarmerie pour assurer la prévention du rassemblement illégal. Je demande le retrait